Monsieur le président,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 Mes chers collègues, par lettre en date du 14 avril, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 18 mai, après-midi et soir, et, éventuellement, du mercredi 19 mai, après-midi, sous réserve de son dépôt et de sa transmission, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. En conséquence, - d'une part, l'examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique et du projet de loi organique modifiant la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est reporté au mercredi 19 mai, après-midi et soir, et, éventuellement, au jeudi 20 mai matin, à l'issue de l'examen des deux propositions de loi déjà inscrites à l'ordre du jour, après-midi et soir d'autre part, l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances est reporté au jeudi 20 mai, à la suite des textes déjà inscrits à l'ordre du jour, et, éventuellement, au vendredi 21 mai, matin et après-midi. Acte est donné de ces demandes. Nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire au mardi 18 mai à 12 heures.

jour, M. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants- République et Territoires, demandent l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de résolution présentée par MM. Alain Richard et Joël Guerriau, en application de l'article 34-1 de la Constitution, en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales. Nous pourrions inscrire ce texte, sous réserve du respect du délai d'information préalable du Gouvernement, en complément de l'ordre du jour du jeudi 6 mai après-midi. Comme il est d'usage lors de l'examen des propositions de résolution, les interventions des orateurs des groupes vaudront explications de vote sur le texte. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Enfin, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, en accord avec le Gouvernement et le groupe Écologiste- Solidarités et territoires, et après consultation de l'ensemble des groupes politiques, le débat sur le thème : « Les enjeux nationaux et internationaux de la future PAC » serait désormais inscrit à l'ordre du jour du mardi 4 mai, le soir et le débat sur le thème : « Contrat de relance et de transition écologique, ne pas confondre vitesse et précipitation » serait désormais inscrit à l'ordre du jour du mercredi 5 mai en dernier point de l'ordre du jour de l'après-midi. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi d'expérimentation visant à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active

je tiens à vous présenter ma position sur le texte que nous examinons. Comme cela a été rappelé lors de la discussion générale, cette proposition de loi est issue des travaux du conseil départemental de l'Allier, lequel est à l'origine de cette initiative et l'a partagée avec l'ensemble des parlementaires du L'objectif est de favoriser le lien entre l'économie et l'insertion en permettant, plus qu'aujourd'hui, le cumul du RSA et d'un salaire un nouveau dispositif. Les départements ont toujours été attentifs à la situation des entreprises et au maintien de l'emploi. Ils sont bien souvent déjà à l'origine de politiques volontaristes et nécessaires qui ont largement structuré les démarches des publics en insertion. cette expérimentation offre un nouveau cadre qui encourage la reprise d'activité des bénéficiaires du RSA, tout en répondant aux besoins des entreprises. Il faut savoir que, dans mon département, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA s'élève à environ 10 000. En parallèle, le nombre d'offres d'emploi est quasiment identique. Ainsi, cette expérimentation aura tout son sens. Le département est un échelon de proximité indispensable. Il finance le RSA, en partie sur ses fonds propres et en partie sur les contributions fournies par l'État.

Ces démarches sont d'autant plus pertinentes qu'elles émanent directement des acteurs de terrain. Pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de loi afin d'accompagner cette initiative et de lui donner toutes ses chances. L'amendement

des actions d'insertion plutôt tournées vers l'insertion professionnelle, parce qu'ils ont besoin d'une formation plus adaptée et d'un accompagnement pour retourner à l'emploi, étant plus loin dans

pour que cette expérimentation puisse être généralisée, avec de gros départements urbains, ceux qui sont au-dessus d'un million d'habitants, des départements intermédiaires, entre 300 000 habitants et un million d'habitants, ou des départements ruraux, de moins de 300 000 habitants. Cette discussion, madame la ministre, doit se tenir avec

quand on est bénéficiaire du RSA, on est déjà dans des dispositifs de minima sociaux depuis un moment : avant le RSA, on a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique

que ce n'est pas l'entreprise qui va « trier » les bénéficiaires du RSA. C'est le travailleur social qui, pour ces publics, est en lien avec le collaborateur de Pôle emploi,

des difficultés à un moment ou un autre ; élargir le dispositif aux publics qui sont peut-être les moins éloignés ne veut pas dire que les plus éloignés n'auront pas leur place. En revanche, je défends l'entreprise, que je connais bien. Pour elle, il n'est pas facile

les personnes volontaires bénéficiaires du revenu de solidarité active privées d'emploi depuis un an ou moins et domiciliées dans les départements participant à l'expérimentation. Le présent amendement vise à apporter une précision et à imposer un nouveau critère pour pouvoir y prétendre : avoir obligatoirement signé en amont un contrat d'engagements réciproques (CER). L'établissement de ce contrat permet l'énumération des engagements réciproques des parties en termes d'insertion professionnelle et formalise la mise en oeuvre du projet d'insertion. Comme pour le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), le CER consacre des droits et obligations qui lient bénéficiaires et collectivités. Il précise, notamment, les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il permet donc d'être sûr de la bonne foi et de la motivation des personnes volontaires pour cette expérimentation. Au niveau national, le taux de contractualisation atteint seulement 52 un chiffre bien trop faible, alors même qu'il s'agit d'une obligation. Lors de l'examen des amendements de séance en commission des affaires sociales, le 14 avril, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement,

la majorité des allocataires. Le CER ne concerne que les bénéficiaires du RSA qui sont orientés vers un organisme autre que Pôle emploi. En effet, les allocataires orientés vers Pôle emploi élaborent, pour leur part, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Par ailleurs, si l'on ne peut que déplorer le

c'est que les travailleurs sociaux qui gèrent son dossier savent qu'il est en mesure de reprendre immédiatement un emploi ; ceux qui sont orientés vers les travailleurs sociaux sont ceux pour lesquels on a décelé un certain nombre

Madame Lubin, vous dites qu'un contrat de travail sera signé avec l'entreprise ; certes, mais les CER, eux, doivent être signés en amont, dès que la personne bénéficiaire du RSA entre dans ce processus d'insertion. Même s'il est satisfait, je maintiens mon amendement, monsieur le

Tous les mois ou tous les deux mois, selon les pratiques, les comités locaux d'insertion se réunissent avec les acteurs représentant les associations, les entreprises, les élus. Et les bénéficiaires qui ne remplissent pas

Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 12, présenté par Mme Lubin,

Il s'agit, par le biais de cette expérimentation, d'encourager une inscription dans l'emploi durable avec le soutien des entreprises, et non de donner une prime aux contrats courts.

l'avis du Gouvernement ?

Le dispositif envisagé dans cette proposition de loi ne garantit en rien que les allocataires du RSA qui en relèveraient auraient plus de chances de s'insérer définitivement à la sortie du dispositif. Je crains également que ce que vous proposez ne soulève un autre sujet, celui de l'effet de seuil à la sortie du dispositif, avec de possibles pertes de revenus,

salaires. Oui, aujourd'hui, il faut relever les salaires de tous ceux qui, gagnant le SMIC, ont du mal à joindre les deux bouts ! J'étais vraiment heureuse de vous entendre tenir ces propos,

qui est de favoriser le retour à l'emploi. Il peut en effet être utile de permettre un coup de pouce, le cumul du RSA et des revenus de l'emploi, pour des durées d'emploi bien plus réduites. J'en veux pour preuve les initiatives lancées par le conseil départemental de Loire-Atlantique,

relatives aux femmes. En France, si les femmes représentent aujourd'hui environ 48 % de la population active, elles sont toujours aussi nombreuses à occuper des emplois précaires : 82 % des salariés à temps partiel et deux tiers des travailleurs pauvres sont des femmes. En dépit de quarante ans de lois sur l'égalité professionnelle, celle-ci n'est toujours pas réalisée. Ce constat appellerait des mesures fortes afin que l'égalité professionnelle ne reste pas un voeu pieux. Pourtant, les dernières réformes du code du travail n'ont fait que fragiliser l'édifice législatif en faveur de l'égalité professionnelle. Le recours de plus en plus massif au temps partiel par les entreprises pénalise en premier lieu les femmes, qui restent les principales variables d'ajustement de l'organisation du temps de travail. 78 % des salariés en temps partiel sont des femmes et 31 % des femmes salariées sont à temps partiel, contre seulement 7 % des hommes. Quant au temps partiel subi, il concerne 32 % des femmes travaillant à temps partiel. Plutôt que de favoriser les mini-boulots de quinze heures par semaine, comme nous y encourage cette proposition de loi, il faudrait davantage encadrer le temps

Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous observons toujours avec attention les propositions qui permettent d'améliorer l'insertion des bénéficiaires de minima sociaux.

il faut bien appeler un chat un chat ! -vivent de ce qu'on veut bien leur donner, il faut qu'ils le méritent en faisant, comme je l'ai entendu ce matin, des travaux d'intérêt général. Je rappelle tout de même que les travaux d'intérêt général sont pour les délinquants ! Je constate aussi que, depuis quelque temps, c'est la fête à la maison ! Il y a peu, on nous a proposé de supprimer les allocations familiales pour ces parents indignes qui ne sont plus capables de s'occuper de leurs enfants.

les plus pauvres de notre société. Nous ne pouvons accepter de casser encore davantage le code du travail avec des sous-contrats à temps partiel de quinze heures.

par le Gouvernement il y a un an et demi et l'association ATD Quart Monde ne siège plus au CESE depuis quelques semaines. C'est regrettable ! Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température ! Nous voterons donc contre ce texte, et nous continuerons, pour notre part, à lutter pour l'amélioration des droits des travailleurs. La parole

que les positions sont divergentes et, parfois, radicalement opposées, mais chacun les a exprimées dans le respect des opinions des uns et des autres ; j'y suis très sensible. Si ce texte est adopté et si nos collègues députés y donnent une suite favorable, c'est l'expérimentation qui nous dira si nous sommes ou non allés dans la bonne direction.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous sommes réunis dans cet hémicycle pour évoquer le CETA (-accord économique et commercial global), ce n'est malheureusement pas sur l'initiative du Gouvernement. Non, chers collègues, c'est le groupe CRCE qui vous y invite, et ce pour la deuxième fois après le débat que nous avons organisé ici même, en novembre 2018, un an après la mise en application provisoire de cet accord ! Depuis trois ans, des parlementaires de presque tous les groupes qui composent cet hémicycle ont demandé au Gouvernement des précisions sur ce traité et sa date de ratification. Nous pensons que le Sénat a été assez patient. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative. Cela étant, je veux que chacun entende une chose en tant que groupe minoritaire et d'opposition, nous n'avons que deux niches par an, c'est-à-dire l'équivalent de quatre textes. Vous avouerez que c'est peu, car, comme vous, mes chers collègues, nous fourmillons d'idées- pas les mêmes, j'en conviens. Pourtant, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de consacrer à ce texte un de nos rares espaces. Nous ne nous résignons pas comme vous à ce déni démocratique constaté et évident. Puisque nous sommes empêchés de débattre par le Gouvernement, le groupe CRCE met son espace à votre disposition avec cette proposition de résolution invitant le Gouvernement à envisager la poursuite de la procédure de ratification du CETA. De nombreux collègues nous ont interpellés sur cette formulation quelque peu alambiquée. Je souhaite vous en expliquer les raisons en toute transparence. Notre proposition a dû être remaniée trois fois avant que le Gouvernement, fort tatillon sur la manière dont nous osions nous adresser à lui, ne daigne l'accepter et en valider la mise à l'ordre du jour dans cette niche parlementaire. Certes, c'est au Gouvernement et non au Parlement que revient l'initiative de la procédure de ratification, et nous savons que le Parlement ne peut pas enjoindre le Gouvernement. Pourtant, avec cette proposition de résolution, nous cherchions non pas à empiéter sur ses pouvoirs, faire respecter nos institutions, la Constitution, le processus démocratique et la compétence du Sénat, qui, je le rappelle, n'est ni optionnelle ni consultative. Il est tout de même assez surprenant, monsieur le ministre, que le Gouvernement, qui bafoue le droit du Parlement, s'insurge lorsque celui-ci ose lui rappeler de respecter notre institution et la Constitution. En somme, non seulement nous ne sommes pas consultés, mais en plus rogne-t-on sur toute proposition que nous faisons.

plutôt que d'ergoter sur sa formulation, de donner directement au bureau du Sénat le calendrier de la procédure de ratification du CETA ! Je rappelle également, puisque cela semble puisque cela semble nécessaire, l'article 53 de notre Constitution, qui dispose que ces traités « ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu d'une loi d'une loi ». La ratification est de fait soumise au vote du Parlement ; un Parlement qui, en France, est bicaméral. En agissant de la sorte, force est de constater que le Gouvernement donne l'impression de considérer que l'avis, les débats et le vote de la Haute Assemblée n'importent guère ; seule compterait donc pour lui l'Assemblée nationale sous la V République ? Le Parlement est sans cesse contourné ou malmené. C'est le révélateur d'une crise plus profonde de nos institutions. Depuis 2017, date à laquelle je suis devenu parlementaire,

l'a rappelé il y a quelques jours, 51 % des textes ont été ratifiés par ordonnance, ce qui est inédit depuis la guerre d'Algérie. doivent ensuite être ratifiées par le Parlement ; la procédure est donc, au bout du compte, deux fois plus longue ... Derrière le prétexte de la recherche d'efficacité ou de rapidité, c'est donc bien le débat au Parlement qui vous contrarie et que vous voulez empêcher. Enfin, alors que nous traversons une crise inédite, avec la covid-19, nous pensons que la démocratie et le débat parlementaire sont une des solutions de la sortie de crise,

qu'une gestion de crise centralisée, concentrée dans les seules mains de l'exécutif, n'est pas gage d'efficacité ni de réussite. Le comble a été atteint quand vous nous avez invités à débattre des mesures à prendre sur le troisième confinement, alors que tout avait été annoncé, la veille, à la télévision, par le Président de la République. Une République dans laquelle le Gouvernement, voire le Président de la République, déciderait seul et où le Parlement validerait tout, sans rien dire, sans discuter, sans critiquer est-elle bien la République que nous voulons ? Selon nous, il n'est pas souhaitable de jouer ainsi avec nos institutions, car cela renforce la défiance de nos concitoyens, qui peuvent légitimement se poser la question si le Gouvernement ne respecte pas la Constitution et les institutions, à quoi sert-il de voter ? En outre, entre l'Union européenne, les citoyens français et la question démocratique, il y a déjà une histoire. Tout le monde se le rappelle, en 2005, après un débat éclairé, populaire et citoyen, le peuple français avait rejeté massivement le traité constitutionnel, finalement imposé par un vote du Parlement, deux ans plus tard. Cette meurtrissure dans le coeur des Français ces derniers, l'idée que l'Union européenne est une instance technocratique, éloignée de leurs préoccupations et antidémocratique. Cela nourrit le fatalisme et le désespoir et explique, en partie, la montée de l'extrême droite partout en Europe. Avec le CETA, ce n'est pas le vote des Français qui n'est pas respecté, c'est celui des sénatrices et des sénateurs qui est empêché. De bout en bout, l'histoire de ce traité pourrait se résumer en un mot opacité ; opacité pendant les sept longues années de négociations et opacité, ensuite, dans sa mise en oeuvre. En effet, cet accord est entré en vigueur de façon provisoire, il y a maintenant plus de trois ans, le 21 septembre 2017, mais c'est un « provisoire » qui dure et qui concerne, tout de même, 90 % du traité, à savoir les compétences exclusives de l'Union européenne. Rien que le principe de cette entrée en application avant que les États membres aient accepté ou non

c'est surtout sur la levée des barrières non tarifaires que nous devrions échanger : remise en cause de nos normes sociales et environnementales ainsi que de nos services publics, mais aussi mise en place de tribunaux d'arbitrages privés, qui permettront, demain, à des entreprises d'attaquer des États au nom du profit du profit ! La crise de la covid-19 a démontré que tout nous invite à repenser le monde différemment, à repenser les échanges, la circulation des marchandises et des capitaux, la relocalisation de nos modes de production ou encore la question de notre souveraineté, notamment alimentaire.

devait être soumis à ratification par le Parlement dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur provisoire. Un an ! Cela fait trois ans que nous attendons !

Il se chuchote, ici ou là, que vous ne l'inscrivez pas à l'ordre du jour du Sénat, parce que vous auriez peur d'un vote contre ; il est vrai que cet accord ne fait pas l'unanimité, et c'est un euphémisme. Néanmoins, pour ma part, je n'ose y croire, car je ne peux imaginer qu'un gouvernement ne soumette au vote des parlementaires que des textes dont il serait certain d'emporter l'adoption et que, en cas de doute, plutôt que d'affronter le débat avec des arguments, il préfère contourner l'obstacle.

nous n'avons pas cherché à lancer, aujourd'hui, un débat sur le CETA lui-même, sur sa pertinence et ses fondements idéologiques, bien que ce débat soit nécessaire. Vous connaissez notre opposition à ce traité, mais nous respectons tous ceux qui y sont Même si nous traversons une pandémie et que les urgences sont nombreuses, cette question traverse la société, comme l'a montré l'exigence, exprimée par la Convention citoyenne pour le climat, d'un moratoire sur ces traités de libre-échange,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Lettonie, le 23 février 2017, puis la Lituanie, le Danemark, Malte, l'Espagne, la Croatie, la Tchéquie, le Portugal, l'Estonie, la Suède, la Finlande, la Roumanie,

En France- pays fondateur de l'Union européenne -, alors même que l'article 53 de la Constitution précise explicitement que le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres, doit ratifier l'accord,

Reste une option : l'oubli volontaire qui arrange. Je m'explique. Pour le Président de la République, le CETA « va dans le bon sens »- ce sont ses mots,

Voilà pourquoi je remercie le groupe CRCE d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette proposition de résolution et de nous obliger à faire un peu d'archéologie, afin de retrouver les positions, sur le

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà trois ans que le CETA est entré en vigueur provisoirement ; voilà pourtant trois ans que le Sénat attend d'avoir à exprimer sa position sur le sujet, lors d'un vote solennel et voilà trois ans que le Gouvernement lui refuse ce droit ... Le CETA divise, vous le savez. Ce ne sont ni l'équilibre global de l'accord ni les relations historiques avec nos compatriotes canadiens qui sont en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le fait de sanctionner, dans chaque accord de libre-échange, toujours les mêmes acteurs : certaines de nos filières agricoles. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à protéger notre agriculture des importations déloyales, qui risquent de nous faire perdre notre souveraineté alimentaire. Ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité politique à tenir des engagements fermes que vous avez pris en matière de respect de nos normes. Or vos réponses peinent à convaincre, car cet accord, on le sait, n'apporte aucune garantie sur la conformité aux normes européennes des produits alimentaires importés. Vous nous rétorquez chaque fois qu'il n'y a aucun problème, que, grâce aux organismes certificateurs et aux limites maximales de résidus prévues dans la réglementation européenne, il n'y a aucun risque et que tout est garanti : ceinture et bretelles ; aucune faille ! Sauf une : personne ne vous croit ... Pour illustrer mon propos, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, au sein de l'Union européenne, un consommateur qui souhaita manger, en quantité, de petites graines de sésame. Pour en retrouver dans son pain, son houmous, ses biscuits, il importa massivement ces graines d'Inde. Mais, tout à coup, en 2020, lors d'un contrôle de routine, des résidus d'une substance strictement interdite en Europe depuis 1991- l'oxyde d'éthylène -furent retrouvés sur ces graines, à des taux mille

car il concernait des produits contenant des graines importées non seulement d'Inde, mais également de nombreux pays dans le monde, et ce depuis 2018 au moins. Comment toutes ces graines avaient-elles pu entrer, comme par magie, en Europe, sans que le problème soit visible, durant tout ce temps ? Premièrement, il n'y avait pas suffisamment de tests aléatoires pour identifier les risques ; comment cela serait-il possible, avec un budget dédié aux contrôles ne dépassant pas, en France, 50 centimes pour 1 000 euros de denrées alimentaires introduites ? Difficile, dès lors, de repérer des dépassements de limites maximales de résidus Deuxièmement, les contrôles douaniers avaient déjà repéré des anomalies sur les résidus de pesticides en provenance d'Inde, puisque 20 % des denrées indiennes aléatoirement contrôlées en 2018 présentaient des anomalies, mais, même quand nous savons, nous ne faisons rien pour inverser la donne. Troisièmement, sur les 1 500 substances actives interdites à l'échelon européen, seules 600 sont effectivement contrôlées. Les importations de denrées dans l'Union européenne sont donc indemnes de 900 substances, car, tout simplement, nous ne les recherchons pas

Si nous ne parvenons pas à contrôler les graines de sésame indiennes, comment pouvez-vous affirmer, monsieur le ministre, que nous serons capables de le faire pour tous les produits canadiens ? Comment pouvez-vous nous assurer, la main sur le coeur, qu'aucune denrée végétale canadienne importée ne méconnaîtra la réglementation européenne, sans même parler des OGM ou des autres substances actives qui sont autorisées au Canada et non en Europe ? Comment pouvez-vous garantir que la viande canadienne respectera nos normes de production, alors que certaines farines animales y sont autorisées et que la traçabilité ne recouvre pas le même champ ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien sûr, le Sénat doit étudier le projet de loi autorisant la ratification du CETA, qui lui a été transmis le 23 juillet 2019. En plus d'être une nécessité constitutionnelle, c'est indissociable de notre démocratie parlementaire. Dans notre pays, le bicamérisme traduit la chance qui est donnée à l'équilibre, à la précision et à la qualité des débats. C'est notre système ; il doit être respecté. La discussion de ce projet de loi au Sénat sera un moment décisif pour la France et pour l'Union européenne. L'enjeu est de taille, dans un processus où l'assentiment des vingt-sept pays de l'Union européenne est nécessaire pour l'application complète de l'accord.

Sur la forme, le retard pris dans le processus de ratification en France est dû à différentes situations, qui ne sont pas toutes le fait du Gouvernement. Ah ? La principale, qui marque malheureusement toujours notre quotidien, est la pandémie mondiale de covid ! Cette crise a bouleversé le calendrier parlementaire et les priorités législatives ; on ne peut pas dire le contraire. Si ! Sur le fond, nous sommes en présence d'un accord dit « de nouvelle génération

à l'affirmation que ces négociations seraient antidémocratiques, revenons sur certains faits. Le mandat de négociation de la Commission européenne a été adopté par les États membres de ses parties ont été rendues publiques. L'accord a ensuite été signé en 2016, notamment par le président du Conseil européen, constitué des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, qui Le chef de l'État français d'alors ne s'y est pas opposé, expliquant que les conditions posées par la France avaient été respectées. Le CETA a ensuite été ratifié par le Parlement européen, élu au suffrage universel direct. Nous sommes conscients que la stratégie commerciale de l'Union européenne est largement perfectible. Après les négociations compliquées avec le Royaume-Uni, la Commission européenne propose de revoir cette stratégie. Des axes cruciaux ont ainsi été dégagés. Deux d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention : la lutte contre la concurrence déloyale et le respect des accords de Paris sur le climat au sein des futurs accords internationaux. Nous ne pouvons que souscrire à ces deux demandes émanant des Européens eux-mêmes. Les valeurs et les intérêts des peuples européens doivent être préservés et défendus. Des craintes concernant le CETA s'expriment. Il faudra des clarifications et des assurances. Surtout, nous devrons rester vigilants par rapport à la mise en oeuvre de cet accord et ne pas faiblir. Nos règles sont différentes dans certains secteurs, notamment en matière alimentaire et agricole. L'harmonisation des normes n'est pas prévue pour tirer ces normes vers le bas, et elle ne doit pas Il est crucial que les règles européennes soient protégées, tout comme nos consommateurs. Pour l'heure, le rapport de 2018 de l'inspection générale des finances, cité dans l'exposé des motifs de cette

En revanche, l'Union enregistre une hausse des exportations de nombreux produits, comme le fromage, dont la France est l'un des principaux producteurs. D'après Eurostat, le volume d'exportation de l'Union européenne vers le Canada a fait un bond de 7 %. Le risque réel, que nous ne pouvons pas ignorer, repose sur le règlement des différends entre autorités publiques et investisseurs. La Commission européenne a travaillé sur ce mécanisme, afin de réduire la possibilité de problèmes à

d'un État membre, simplement parce que ces règles entraveraient son commerce. Enfin- j'en terminerai par là -, le 25 mars dernier, le comité conjoint de l'accord commercial entre a rendu des conclusions sur le volet économique du CETA. Celui-ci aurait des effets positifs dans la pandémie que nous traversons. Ainsi, pour le moment, il semble que l'accord apporte plus de points positifs à l'Union européenne qu'au Canada, mais son application n'en est qu'à son début. Nous entendons les craintes et nous en partageons certaines. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants se tient prêt à avoir, au moment voulu, un débat constructif et pertinent sur le projet de loi autorisant la ratification du CETA. avant cela, nos forces devraient peut-être se concentrer sur la gestion de la pandémie et sur la préparation de notre sortie de crise. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.

Voilà bientôt deux ans que l'Assemblée nationale a adopté le texte, et nous attendons toujours que vous daigniez soumettre au Sénat le projet de loi autorisant la ratification de cet accord. Pour imposer un rythme de navette effréné à l'examen de textes électoralistes saccageant la République et instaurant un État policier, il y a du monde de la Constitution et nous consulter sur des mesures déjà actées par le Président de la République, il y a encore du monde ; mais, pour soumettre un accord international à la ratification, de valeur constitutionnelle, de la chambre haute, là, il n'y a plus personne Le Gouvernement ne cesse de nous assurer du respect qu'il a pour notre chambre- le Premier ministre l'a fait, hier encore, à cette tribune -, mais, comme le disait le poète Pierre Reverdy, « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ».

notre endroit. De quoi le Gouvernement a-t-il peur ? Que le Sénat rejette le CETA ? De remettre dans l'actualité un sujet totalement anachronique, un accord du XX siècle, un traité du monde d'avant le covid, un symbole de la mondialisation qui paupérise les peuples et détruit l'environnement ? Ou bien les deux à la fois ? Nous pouvons comprendre cette peur. Alors que la crise a mis à nu des failles béantes de la mondialisation, alors qu'elle a mis en lumière notre besoin criant de résilience et de souveraineté, le CETA ressemble plus que jamais au sparadrap du capitaine Haddock ... Nos agriculteurs ne s'en sortent plus. Lactalis veut supprimer, sur ses bouteilles, l'indication de provenance du lait ; le pauvre ministre de l'agriculture en perd ses bras, et vous voulez continuer à l'affliger Le Canada autorise les farines animales et certains OGM ; la concurrence internationale tire les prix vers le bas et réduit, comme une peau de chagrin, le revenu des agriculteurs nos normes sociales et environnementales sont piétinées au profit des multinationales, dont les pouvoirs sont élargis au point d'empêcher les États de légiférer pour protéger les peuples et la planète. Donner encore davantage de pouvoir aux intérêts privés au détriment de l'intérêt général, est-ce vraiment là votre vision du monde, monsieur le ministre ? Alors que l'Assemblée nationale examine le projet de loi Climat, qui demeure très en deçà des engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, vous faites un énième pied de nez à la Convention citoyenne

le « en même temps » fait des noeuds au cerveau, même aux intelligences supérieures. Cet aveuglement vous empêche de concentrer vos efforts pour corriger les fragilités du pays relocaliser la production économique, notamment agricole ; protéger notre économie, tout particulièrement nos agriculteurs, de la concurrence déloyale du marché renforcer la puissance publique face aux intérêts privés prédateurs ; engager la transition écologique, notamment agroécologique ; protéger les emplois ainsi que les salaires et instaurer un revenu paysan digne de ce nom développer une économie de circuits courts et de vente directe, loin des multinationales agronomiques, qui exploitent les agriculteurs et sont les principales responsables de la plus grave et de la plus morbide épidémie qui touche la planète : l'obésité. S'il était un exemple de l'hypocrisie totale de votre politique faussement écologique, le voilà sous nos yeux. Le « » a de beaux jours devant lui Au moins, en matière de démocratie, les choses sont claires. Emmanuel Macron pense que la France a besoin d'un monarque, et son mépris du Parlement, de la Convention citoyenne pour le climat, des syndicats agricoles, des ONG et du peuple ne surprend personne. Ce qui est nouveau, c'est que cette soif de pouvoir absolu ne parvient même pas à respecter le cadre et l'usage quasi monarchique de la Constitution de la V République. Comment voulez-vous que les Français vous fassent à nouveau confiance en 2022 ? Le groupe écologiste votera, naturellement et des deux mains, en faveur de cette proposition de résolution. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

a été signé avec le Canada. Ce traité a été approuvé par le Parlement européen en 2017 et ratifié par le Sénat canadien la même année.

on peut citer la décision du Conseil constitutionnel déclarant le CETA conforme à la Constitution et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, que notre collègue Colette Mélot a citée.

le flux d'importation de viande bovine entre le Canada et l'Union européenne est très faible. Ce n'est pas un cas de force majeure. Le Canada a ouvert ses marchés publics dans les secteurs où l'expertise française est reconnue. Les effets positifs de la mise en oeuvre du CETA militent en faveur de la poursuite du processus de ratification.

Parmi les problèmes qui demeurent figurent les modalités d'octroi des contingents d'accès au marché canadien des fromages, lequel est important pour la France, l'accès au marché des vins et spiritueux au Canada, lui aussi important pour la France, et la protection effective des indications géographiques de tous nos produits. Il est par ailleurs nécessaire de poursuivre l'évaluation du CETA au regard de l'accord de Paris. Le Président de la République s'est engagé : il a déclaré n'avoir « aucun tabou » et être prêt à abandonner le CETA « si l'évaluation montre qu'il n'est pas conforme à la trajectoire de l'accord de Paris

cela est prévu depuis 2016 : le CETA étant « mixte », il requiert l'unanimité et doit par conséquent être ratifié par le Parlement de chacun des États membres de l'Union européenne. Or il n'y a eu qu'un seul vote, à l'Assemblée nationale, en juillet 2019

pour évaluer les enjeux environnementaux et sanitaires du CETA, avaient conduit le Gouvernement à élaborer, la même année, un plan d'action pour sa mise en oeuvre. Celui-ci contenait des engagements ambitieux sur le rôle du Parlement. C'est sans doute oublié ! Les enjeux ne sont pas anodins. Le CETA, document de plus de 2 000 pages, comprend des mesures d'accès réciproque des parties à leurs marchés. Au-delà de la baisse ou de la levée des droits de douane, il est question de la réduction des obstacles non tarifaires, de l'assouplissement de l'accès aux marchés publics ou encore d'harmonisation des règles en matière de propriété intellectuelle. Depuis 2017, les accords de libre-échange dits « de nouvelle génération » ne se limitent pas à des dispositions de nature commerciale relevant exclusivement de la compétence de l'Union européenne. Ces accords intègrent également de nombreuses clauses portant notamment sur l'investissement, la coopération réglementaire ou le développement durable, certaines de ces clauses relevant de la compétence des États membres. Autre problème soulevé par cette absence de ratification : l'accord de partenariat stratégique (APS) n'est lui non plus toujours pas promulgué par le Canada, bien qu'il ait été approuvé en 2017 par le Parlement européen, en même temps que le CETA. Le gouvernement canadien attend la fin du processus de ratification des États membres de l'Union européenne. On parle peu de cet accord, qui n'a pas cristallisé l'opposition en 2016. Pourtant, il est majeur, car il rassemble le volet politique. Il aborde les valeurs partagées, par exemple les questions de développement durable, la bonne gouvernance fiscale et le rôle de l'OMC. La proposition de résolution de notre collègue Fabien Gay que nous examinons aujourd'hui est primordiale : elle vise à demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat du projet de loi de ratification du CETA. Nous le savons, une partie de notre assemblée va s'y opposer.

La Convention citoyenne pour le climat a d'ailleurs demandé au Gouvernement de dénoncer l'application provisoire du texte de libre-échange tant que l'accord de Paris n'y serait pas intégré, alors qu'il figure au sein de l'APS. Cet accord comporte des incohérences dont il nous faut débattre. Nous devons nous exprimer à ce sujet, poser les questions qui fâchent, comme son impact réel sur notre agriculture. Si les chiffres fournis témoignent d'une hausse des exportations européennes globales vers le Canada et les États-Unis de 15 % en 2018, nous devons objectiver ces données en 2021, plus particulièrement pour l'agriculture, qui paie souvent le prix cher de ces accords internationaux. N'oublions pas, chers collègues, que se dessine le Mercosur, sur le même modèle que le CETA. La gouvernance de l'Union européenne montre bien ses limites politiques : la Commission décide, les accords sont appliqués et les Parlements des États membres ratifient plus tard ... ou pas. Nos agriculteurs sont toujours sacrifiés sur l'autel d'accords internationaux qui bénéficient, certes, à d'autres secteurs français. Il est de notre devoir moral d'imposer ce débat au Sénat. Même si le résultat ne correspond pas à la ligne directrice de la Commission européenne, le groupe du RDSE votera pour cette proposition

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 23 juillet 2019, l'Assemblée nationale a examiné en urgence, en fin de session extraordinaire, le projet de loi de ratification du CETA. Deux ans plus tard, quatre ans après sa signature, ce texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Pourquoi un tel déni ? Comment justifier le silence du Gouvernement qui accompagne cette non-inscription ? Le Gouvernement a-t-il l'intention de contourner définitivement le vote de notre chambre en jouant la carte de l'application provisoire indéfinie, puisque aucun délai légal de ratification ne s'impose à la France ?

Après tout, pourquoi s'embarrasser d'un vote du Sénat qui pourrait être défavorable et d'un retour incertain devant l'Assemblée nationale ? C'est le raisonnement que semble faire le Gouvernement. Est-ce acceptable ? À l'évidence, non, et je veux citer les raisons majeures qui appellent cette discussion dans notre assemblée. La première est l'impératif démocratique, largement souligné par notre collègue Fabien Gay. Les chefs d'État européens et la Commission européenne ont malheureusement pris de fâcheuses habitudes de contournement démocratique des parlements comme des mobilisations citoyennes. Dès lors, comment s'étonner du désaveu populaire ? La deuxième raison tient évidemment au contenu du CETA. Cet accord est d'une très grande importance. Il s'inscrit dans la lignée d'une libéralisation effrénée des échanges, qui se paie en abaissement des normes, en délocalisations industrielles massives, en dépendance accrue de notre pays dans des secteurs essentiels, comme l'agriculture, mais aussi la pharmacie et le médicament ou le numérique. Continuer à appliquer des accords comme celui du CETA sans ratification ni évaluation n'est pas responsable. La révolution écologique, nous le savons, n'est plus une option. Cependant, elle soulève d'énormes défis de transition. La relocalisation de nos productions et un renforcement de nos services publics sont indispensables pour répondre à la crise que nous traversons. Dans ces conditions, l'évitement de l'exécutif sur ce sujet révèle un embarras manifeste et problématique. D'ailleurs, le Président de la République avait déjà sorti son joker pour évincer la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui s'opposait au CETA Il est pourtant devenu évident que la mondialisation financière sans garde-fous, tournée vers la compétitivité à tout prix et bâtie sur le dogme de la concurrence libre et non faussée est, dans bien des domaines, responsable de l'incapacité de nombreux États, dont la France, à faire face aux nouveaux défis d'avenir : la réduction des inégalités, le climat, la pandémie ...- il y en a bien d'autres. Les accords de libre-échange comme le CETA et, demain, le Mercosur nous désarment face aux défis qui s'aiguisent, au lieu de reconstruire les conditions productives, sociales et environnementales pour les relever. Le CETA ouvre la voie à une nouvelle génération d'accords de libre-échange qui s'étend désormais aux barrières non tarifaires et qui touche tous les domaines : l'environnement, l'agriculture, les protections sociales, les réglementations sanitaires, les investissements, les marchés publics. Il s'agit de tirer toujours vers le bas les normes sociales et environnementales. La commission Schubert, qui a conduit une analyse indépendante du CETA, a souligné le « manque d'ambition » environnementale du traité. De fait, le CETA continuera d'entraîner une augmentation des émissions liées au fret transatlantique, l'encouragement de la concurrence des pratiques d'agriculture les plus intensives, contraires aux objectifs affichés par l'Europe, la mise en berne des normes protectrices du climat et de l'environnement. J'ajoute enfin qu'aux dangers déjà évidents s'additionnent désormais ceux que révèle dramatiquement la pandémie. Nous avons besoin de coopération et non d'exacerbation de la concurrence. Nous avons besoin de reconquérir de la souveraineté, en alliant la protection de normes nationales exigeantes et de coopérations fondées sur la promotion de biens communs, et non de productions rentables à tout prix, quoi qu'il en coûte. Le débat sur les vaccins et la libération des brevets en est un bel exemple. L'OMC discute d'ailleurs actuellement de nouvelles règles permettant de mieux relever ces défis pour toute la planète et pour toute l'humanité. Est-ce le moment de pousser dans ce sens ou, au contraire, de laisser prospérer les logiques moins-disantes et ultraconcurrentielles d'accords comme le CETA ? c'est en tout cas le moment, quelles qu'aient été au départ nos positions sur le CETA et quelles qu'elles soient encore aujourd'hui, d'avoir ensemble un débat approfondi, respectant les prérogatives du Parlement. Ensemble, nous pouvons demander au Gouvernement de répondre à cette exigence en votant la proposition de résolution que le groupe CRCE vous soumet aujourd'hui.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cette proposition de résolution, nos collègues du groupe CRCE nous invitent à rappeler au Gouvernement qu'il serait temps de mener à son terme la procédure de ratification du CETA. En France, celui-ci a été voté par 266 députés en juillet 2019, mais, depuis, il n'a toujours pas été soumis à l'approbation du Sénat. Nous sommes impatients, monsieur le ministre, d'en connaître les motifs, car nous ne pouvons imaginer que vous vous satisfaisiez de la situation actuelle, avec un traité en vigueur seulement partiellement et pour et pour une durée indéterminée. Par ses tergiversations, le Gouvernement donne aujourd'hui le sentiment de craindre le Parlement, comme s'il n'était pas prêt à assumer les conséquences de ce traité dans les territoires. Pour beaucoup de centristes, qui pensent que l'avenir de la France passe par une Europe plus démocratique, plus unie et plus forte, la procédure choisie, qui écarte le référendum et relègue les parlements nationaux à des chambres d'enregistrement, porte déjà en elle-même préjudice à l'ambition européenne. Par son défaut de transparence, elle détériore la confiance des citoyens en leurs institutions. Au-delà de la légitime demande de démocratie et de respect des procédures de ratification qui vous est il y a une dimension plus pragmatique et plus politique, qui plaide pour un débat rapide au Sénat et sur laquelle, vous l'avez compris, nous aimerions vous entendre, monsieur le ministre s'agit de la pertinence de ce traité dit « de deuxième génération », mais finalement déjà dépassé dans un monde post-covid et d'urgence climatique. Depuis un an, en effet, nous mesurons chaque jour combien la souveraineté économique, alimentaire, numérique médicale, l'urgence climatique et le bilan carbone sont devenus de nouvelles priorités. Ces réalités n'avaient pas la même acuité voilà quinze ans, lors des négociations du CETA. Aujourd'hui, ces défis sont devant nous, et nous sommes en droit de nous interroger est-il bien cohérent de supprimer des droits de douane, alors que, dans le même temps, nous envisageons d'imposer des taxes carbone aux frontières ? Alors que la France et l'Europe imposent à leur production des écoschémas, des circuits courts de la ferme à la fourchette, un, des analyses du cycle de vie, des normes RSE, une lutte contre la déforestation, devons-nous continuer à laisser entrer des produits qui ne répondent pas à ces critères pour respecter les contreparties de traités ? Très bonne question ! À l'heure de l'urgence climatique, le commerce international peut-il encore consister à importer ce que nous ne voulons pas pour vendre ce que nous voulons exporter ? Le moment est-il bien choisi pour lever tout obstacle aux investissements étrangers, alors que l'enjeu de souveraineté économique n'a jamais été aussi stratégique ? Faut-il soumettre nos États aux arbitrages de tribunaux spécifiques visant à protéger « les attentes légitimes des investisseurs internationaux », et non les intérêts des citoyens, à l'heure où l'on plaide pour plus de régulation et pour un retour des États, notamment dans les secteurs numérique, alimentaire, de la santé et de l'environnement ? Toutes ces interrogations pressantes, auxquelles nous n'avons pas encore de réponses, se heurtent non pas au principe des échanges internationaux, mais aux modalités de ce traité. Elles justifient un débat urgent, que vous ne pouvez ni éluder ni repousser. L'avenir d'un projet européen crédible et d'un commerce ouvert ne se fera pas en occultant les questionnements des parlements nationaux ni même en se contentant de regarder dans le rétroviseur les bilans chiffrés de ces trois dernières années. Ces impératifs nouveaux, qui ont surgi en quelques mois, modifient en profondeur et dans la durée les réalités économiques, commerciales et sociétales à venir. Ils nous obligent à nous adapter, car, nous le savons tous, gouverner, c'est prévoir, d'autant qu'ils s'inscrivent dans l'urgence : l'urgence de neutraliser les changements climatiques, l'urgence de la relance économique et de l'emploi dans les territoires, l'urgence de faire renaître l'espoir chez nos concitoyens. Par respect pour les peuples et pour le pouvoir de représentation qu'ils ont confié au Parlement, par respect pour l'Europe et pour la procédure de ratification choisie, pour la cohérence des politiques publiques et la résilience de nos économies, le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de résolution.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux à mon tour remercier nos collègues du groupe CRCE de leur initiative. Voilà effectivement vingt et un mois que l'Assemblée nationale a voté, à une courte majorité, la ratification du CETA, accord mixte conclu entre l'Union européenne et le Canada qui nécessite la ratification des États membres. Voilà vingt et un mois que nous attendons que le Gouvernement l'inscrive à l'ordre du jour du Sénat et trois ans et demi que cet accord dit « de nouvelle génération » systémique vit sous sa forme provisoire, créant un précédent fâcheux. mon collègue Rachid Temal l'a exprimé justement, nous vivons là un déni et une aberration démocratiques. C'est une mauvaise manière faite au Sénat, mais c'est surtout une manière qui renforce encore la défiance de nos concitoyens à l'égard de ces accords commerciaux aujourd'hui dépassés. dépassés, parce que le monde a changé. La mondialisation libérale et l'accélération des échanges ont, certes, généré de la croissance et permis de développer de nouveaux secteurs, mais elles se sont aussi malheureusement traduites par un accroissement des inégalités territoriales et sociales ainsi que par la destruction de pans entiers de nos économies, laissant des millions de travailleurs européens sur le carreau, sans parler de l'exploitation des travailleurs de nombreux pays du tiers-monde, sous-traitants des multinationales qui nous offrent des produits à bas prix. dépassés, parce que la mutation numérique de nos économies a ouvert de nouveaux espaces de croissance, mais aussi de dérégulation, permettant à des multinationales de dicter leur loi, d'accumuler les profits et d'échapper à l'impôt. dépassés par l'accélération du changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation de l'environnement, qui mettent en péril l'avenir de l'humanité et interrogent nos modèles de développement. Enfin, ces accords sont dépassés par l'essor de la Chine, lequel change fondamentalement l'ordre économique et politique mondial, bouleversant concurrence et gouvernance. l'accord entre la Chine et les quatorze pays de la zone indopacifique conclu en novembre dernier dans la région la plus dynamique du monde illustre le déplacement du centre de gravité dans les rapports de force mondiaux et l'accélération de la régionalisation des marchés. La pandémie de la covid-19 a mis en lumière ces phénomènes en exacerbant les tensions et a permis une prise de conscience accélérée de leurs conséquences économiques et sociales et de leur incidence en matière de dépendance stratégique. Face à cette situation, l'Union européenne n'a d'autre choix que de redéfinir ses relations internationales et ses échanges commerciaux, de nous protéger sans nous isoler ni nous replier. replier. Elle doit se servir de sa position d'acteur commercial majeur pour défendre un modèle de développement commercial équitable et durable et ne pas se trouver marginalisée dans la bataille politique, stratégique et commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. L'Union européenne doit être motrice pour réformer l'Organisation mondiale du commerce, restaurer le multilatéralisme, redéfinir des règles communes et installer de nouvelles instances d'arbitrage. Nous devons porter à l'échelle internationale un niveau d'exigence élevé et promouvoir les normes et standards européens, tout en révisant ceux-ci à la hausse. Les accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux doivent dorénavant inclure la lutte contre le dérèglement climatique, la défense de nos normes sanitaires et environnementales, le respect des droits de l'homme, la protection des travailleurs et un devoir de vigilance de nos entreprises et de celles des pays tiers, qui devront respecter des exigences sociales élevées. La Commission européenne a récemment présenté sa feuille de route pour redéfinir sa politique commerciale. Si celle-ci ouvre des perspectives positives, elle ne va pas au bout de la démarche. La redéfinition de la finalité de ces accords ne tire pas toutes les leçons des interrogations et des doutes qui traversent les opinions publiques européennes. Si, sous l'impulsion de la France, lors du quinquennat précédent, des progrès ont été réalisés sur la transparence des négociations, il faut aller plus loin et permettre un débat démocratique pour s'assurer que la politique commerciale est au service du bien commun. La Commission évoque la réforme de l'OMC et de plus grandes exigences dans les différents domaines que j'ai cités, mais l'objectif d'une « autonomie stratégique ouverte » laisse perplexe. Elle ne remet pas en cause le dogme libéral au bénéfice du juste échange et ne prévoit pas de stratégie de relocalisation et de rapatriement des chaînes de valeur. question de la nature juridique de ces accords qui est posée. Celle de la compétence exclusive de la Commission européenne, celle de la durée des mandats de négociation- vingt ans pour le Mercosur ... -, celle, pour les rares accords mixtes, de l'absence de date butoir de ratification

Nous avons besoin aujourd'hui d'une pause, d'un moratoire sur les négociations et d'une redéfinition démocratique des critères environnementaux, sociaux, fiscaux et de droits humains, qui doivent être au coeur des échanges. être ambitieux et remettre les accords commerciaux au service d'un modèle de développement équitable et durable qui serve d'outil au bénéfice d'une Europe géopolitique. La France, monsieur le ministre, aura, à ce titre, une responsabilité particulière, puisque la présidence française devra faire aboutir les négociations sur la nouvelle stratégie commerciale entre les États membres. Les conditions seront alors réunies pour clarifier en premier lieu au niveau national les termes du débat autour de la politique commerciale commune. C'est à l'aune de ces remarques que, le jour venu, si le Gouvernement en décide, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain se prononcera sur le CETA. Nous espérons que cette inscription à l'ordre du jour du Sénat viendra très vite, raison pour laquelle nous voterons la proposition de résolution du groupe CRCE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, signé le 30 octobre 2016 par le Canada et l'Union européenne et ses États membres, le CETA a été approuvé par le Parlement européen en février 2017. est un accord commercial bilatéral de libre-échange « de nouvelle génération ». Il ne se contente pas de réduire les seuls droits de douane, mais tente de diminuer toutes les entraves au commerce. Ainsi, outre la baisse des droits de douane, le CETA prévoit la protection des appellations d'origine contrôlée européennes, l'assouplissement de la mobilité professionnelle ou encore l'ouverture des marchés publics canadiens. Le CETA, c'est aussi la modification de quotas, dont l'augmentation des importations de viande canadienne vers l'Europe. Certaines de ses dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne et d'autres des États membres, ce qui implique sa ratification par les parlements des vingt-sept États membres. Quatre ans plus tard, seuls treize pays européens l'ont ratifié.

a néanmoins autorisé l'application provisoire des dispositions du CETA relevant de la compétence exclusive de l'Union. de l'accord sont entrées en vigueur le 21 septembre 2017, sans que le Parlement français se soit jamais prononcé. En France, le processus de ratification n'a été amorcé qu'à l'été 2019, avec le dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi de ratification. Le 23 juillet, après plusieurs jours d'âpres débats et l'opposition marquée du monde agricole, ce texte a finalement été adopté à une courte majorité, par 266 voix contre 213.

Avec mes collègues de la commission des affaires économiques, nous étions prêts. Nous avions même désigné notre rapporteur pour avis. Deux ans après sa ratification par les députés, quatre ans après son entrée en vigueur, le Sénat n'a toujours pas eu à se prononcer. Qu'attend-on ? République a rejeté l'appel de la Convention citoyenne pour le climat à renégocier le CETA. A-t-il peur que nous n'imitions nos collègues chypriotes ? Le Sénat doit pouvoir débattre et s'exprimer sur cet accord, qui peut interroger en matière de sécurité sanitaire, de qualité des produits importés, mais aussi de préservation du modèle agricole français. Le Sénat doit pouvoir débattre et s'exprimer sur l'opportunité d'un tel accord, dont les négociations ont débuté en 2009, dans une société qui n'avait pas pleinement conscience des enjeux climatiques. Le débat est d'autant plus indispensable qu'un audit de la Commission européenne de mai 2020 a confirmé certaines craintes traçabilité défaillante du bétail, conflits d'intérêts potentiels des vétérinaires chargés d'évaluer le respect des règles sanitaires La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui invite le Gouvernement à permettre ce débat. Nous partageons ce souhait. Une fois n'est pas coutume, je tiens à féliciter nos collègues du groupe CRCE de leur initiative. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant près de deux ans, l'Assemblée nationale ratifiait l'accord économique et commercial global, dit CETA. Cet accord entre l'Union européenne et le Canada organise les aspects tarifaires des échanges de biens et de services, la régulation des investissements et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe CRCE nous propose d'adopter une résolution invitant le Gouvernement à envisager la poursuite du processus parlementaire de ratification du CETA. Nous sommes favorables à cette démarche. Elle offrirait au Sénat l'opportunité d'approuver à son tour cet accord historique de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Peut-être pas ! Approuvé par l'Union européenne, le CETA est mis en oeuvre depuis plus de quatre ans et présente déjà des résultats très positifs pour la France. Je vais y revenir.

En économie, c'est pareil. La lecture de l'exposé des motifs de leur proposition de résolution le démontre : le libre-échange, décidément, ça ne passe pas, serait, selon eux, « à l'origine d'une " mondialisation malheureuse " pour les peuples ». Leur document prétend que le CETA répond aux seuls intérêts des multinationales. C'est faux ! Sur les 10 000 entreprises françaises qui exportent, 8 000 sont des PME. Je ne dispose pas du temps nécessaire ... Heureusement ! ... pour pointer toutes les approximations, les exagérations ou les nombreuses élucubrations offensantes sur les réglementations canadiennes dans l'exposé des motifs. Ces propos relèvent du « Canada », et je le regrette. Si cet accord de libre-échange non ratifié est déjà entré en vigueur provisoirement, c'est parce que plus de 90 % des dispositions relèvent des compétences exclusives de l'Union européenne. ! En fait, ce qui irrite profondément le groupe CRCE, comme d'autres, c'est tout simplement que l'Union européenne fonctionne- et cela n'est pas nouveau ! Les faits sont têtus l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et l'Union européenne s'avère déjà très bénéfique pour la France. Nos exportations ont progressé de 24 % dans les trois premières années : 63 % pour les fromages, 96 % pour les produits de boulangerie, 16 % pour les vins et boissons et plus de 30 % pour les cosmétiques, le textile et l'habillement. C'est le monde des Bisounours ! Grâce au CETA, nos entreprises, multinationales ou TPE-PME, peuvent accéder pleinement aux marchés publics fédéraux canadiens, bien au-delà des règles auparavant en vigueur dans le cadre de l'OMC. On observe déjà de nombreux succès : EDF avec le développement de parcs éoliens en Alberta ou encore Vinci avec la construction d'une usine de traitement des eaux en Colombie-Britannique ou d'une autoroute en Alberta. Pour Pierre Touzel, conseiller des Français de l'étranger à Vancouver, le CETA est une chance inouïe de mettre l'Europe au centre du jeu dans l'Ouest canadien, qui a un fort tropisme pour l'Asie. De son côté, Marc Albert Cormier, élu de Toronto, témoigne que nos compatriotes de l'Ontario accèdent désormais à des produits issus de l'agroalimentaire français à des coûts abordables dans les grandes surfaces et magasins spécialisés et que nombre d'entre eux bénéficient également de l'accord dans le cadre de leur emploi. François Lubrina, élu de Montréal, célèbre des succès remportés dans sa ville par Vinci pour le tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine ou Alstom avec le contrat du métro léger. Quand j'écoute nos élus du Canada, je réalise que le CETA s'affirme comme un accélérateur de croissance et de création d'emplois. Il permet aussi d'offrir le mieux-disant au consommateur en termes de normes et de qualité, car le Canadien

monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'ont souligné plusieurs orateurs, le CETA est de nature mixte : une large partie de l'accord, sur le volet commercial, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, en application de l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais une autre partie, relative relative au volet « investissements », relève des compétences partagées entre l'Union et les États membres. À ce titre, cet accord doit être ratifié par les États membres et, donc, en France par le Parlement. C'est cette compétence exclusive de l'Union sur une partie du CETA qui a permis son entrée en vigueur à titre provisoire, à partir du 21 septembre 2017. Il n'y a pas d'ambiguïté quant à la portée du processus de ratification de cet accord par les parlements nationaux. Ils ne sont pas saisis d'un morceau de texte, mais bien de l'ensemble. Si le processus de ratification échoue dans l'un des États membres, l'accord ne pourra pas continuer à s'appliquer. Lorsqu'il a autorisé la signature de l'accord, le Conseil a en effet précisé la portée de l'application provisoire et adopté une déclaration, inscrite au procès-verbal, affirmant que, si la ratification de l'accord économique et commercial global avec le Canada échoue de façon définitive en raison d'une décision prononcée par une Cour constitutionnelle, ou à la suite de l'aboutissement d'un autre processus constitutionnel et d'une notification officielle par le gouvernement de l'État concerné, l'application provisoire devra être et sera dénoncée ». Encore faut-il que les parlements puissent se prononcer. Et c'est là le coeur de notre débat. Le projet de loi autorisant la ratification de cet accord a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2019, le Gouvernement engageant au même moment la procédure accélérée. De fait, la procédure a été rapide à l'Assemblée nationale, puisque le projet de loi y a été adopté le 23 juillet suivant, à une courte majorité. Depuis lors, plus rien Le Gouvernement oublie méthodiquement d'inscrire ce projet de loi à l'ordre du jour du Sénat, empêchant ainsi la poursuite du processus de ratification. Monsieur le ministre, seriez-vous gêné ? Et, dans ce cas, pourquoi ? Les services de la direction générale du Trésor et du Secrétariat général des affaires européennes, que j'ai interrogés récemment, m'ont affirmé que l'application provisoire du CETA est bénéfique pour la France. Douteriez-vous de vos données ou de votre capacité de conviction ? Sinon, pourquoi refuser la reprise du processus de ratification ? La ratification n'est pas une option, la démocratie n'est jamais une option. Un débat exigeant est toujours plus utile que des tentatives de contournement qui alimentent les suspicions et les rancoeurs. Il ne faut pas se le cacher : oui, le CETA est contesté par certaines filières, notamment la filière bovine, évoquée par mon collègue Laurent Duplomb. Oui, la Commission européenne a pu paraître, par le passé, trop naïve et trop lente lorsqu'il s'agissait de protéger les entreprises européennes face aux pratiques déloyales de certains États. Premier importateur et exportateur mondial, premier partenaire commercial de soixante-quatorze pays dans le monde, l'Union européenne est assurément une puissance commerciale. Pourtant, elle n'en a pas suffisamment tiré les conséquences politiques par le passé. Elle n'a pas suffisamment exploité ses atouts et n'a pas été assez vigilante concernant le respect de la mise en oeuvre des accords conclus. Ces faiblesses semblent en voie d'être corrigées. Le titre de la communication, présentée le 18 février dernier par la Commission européenne, pourrait nous le faire penser Oui, il faut assurer un meilleur suivi de la mise en oeuvre des accords et lutter avec fermeté contre les pratiques déloyales. Oui, la politique commerciale de l'Union doit venir en appui de ses intérêts géopolitiques et doit contribuer à l'affirmation de l'autonomie stratégique de l'Union. Ouvert ne veut pas dire naïf. Je souscris également à l'approche consistant à intégrer davantage la politique commerciale et les politiques intérieures de l'Union, en particulier la politique de la concurrence et la politique industrielle. Je l'ai encore dit la semaine dernière En conclusion de sa communication, la Commission européenne souligne vouloir « favoriser un débat éclairé sur la politique commerciale » en approfondissant les contacts qu'elle entretient avec la société civile et les partenaires sociaux, mais sans mentionner les parlements nationaux. Monsieur le ministre, le Parlement n'est pas l'adversaire du Gouvernement ni de la Commission sur ces sujets commerciaux. L'adversaire, c'est la méfiance, voire la défiance, qui peut s'installer chez nos concitoyens. Nous pouvons vous aider à la réduire si nous sommes correctement informés et associés. Alors, aidez-nous à le faire et poursuivons le processus de ratification.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, Jean-Yves Le Drian est en Inde.

CETA. Je voudrais tout d'abord revenir sur ce processus de ratification. Comme vous l'avez souligné, le CETA est un accord mixte dont la majorité des dispositions relève de la compétence exclusive de l'Union Il en comprend d'autres qui relèvent d'une compétence européenne, mais exercée de manière partagée entre l'Union et ses États membres. Certaines dispositions consacrées à la protection des investissements relèvent de cette compétence dite mixte. C'est donc ce premier volet qui justifie la ratification par les parlements des vingt-sept États membres, dont la France, conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution. Comme vous le savez, le projet de loi autorisant le Gouvernement à ratifier l'accord a été approuvé par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2019. Le Sénat

Cette application provisoire ne remet pas en cause les compétences du Parlement ni la légitimité démocratique de cet accord, et ce pour trois raisons : d'abord, l'application à titre provisoire ne concerne que les dispositions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union ensuite, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'application provisoire est conforme à notre Constitution dans sa décision du 31 juillet 2017 ; enfin, l'application provisoire n'a été autorisée par le Conseil de l'Union qu'à la suite de l'approbation de l'accord par le Parlement européen, le 15 février 2017. Ce régime d'application provisoire est donc prévu par le droit international. Un an ! L'application provisoire du CETA nous permet également de suivre très précisément les effets économiques, sanitaires, environnementaux et climatiques de l'accord, conformément au plan d'action mis en place par le Gouvernement dès 2017 et dont nous rendons compte au Parlement de manière régulière. Là encore, une nouvelle fois, je suis à la disposition du Sénat.

avec une hausse de 24 % de nos exportations et une balance commerciale positive pour la France d'un montant record de 650 millions d'euros en 2019. En 2018, notre excédent

Prenons l'exemple des produits agricoles, soit notre premier poste d'exportation : grâce au CETA, ce secteur bénéficie d'importantes baisses de droits de douane canadiens et certaines de nos indications géographiques

IGP françaises sont protégées au Canada. Ainsi, en 2020, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, le vin demeure le premier produit exporté au Canada, à hauteur de 391 millions d'euros, au même niveau qu'en 2019.

peuvent être exportés vers l'Union européenne et entrer sur le marché intérieur et, donc, en France. Le CETA, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à l'instar de tous les accords commerciaux,

Avec Julien Denormandie, nous avons interpellé la Commission européenne lorsqu'elle a publié un rapport pointant des marges de progression dans le système canadien de traçabilité de la viande bovine pour lui demander de travailler avec Ottawa à rehausser le niveau d'exigence canadien. Je suis également intervenu en personne auprès de mon homologue canadienne pour souligner l'importance de cette

Nous avons demandé à la Commission européenne d'y porter une attention particulière dans le cadre de la révision de la politique commerciale de l'Union. Vous pouvez compter sur ma pleine mobilisation pour continuer à défendre cette position à Bruxelles. Par ailleurs, et d'une façon générale, je vous rappelle que la France soutient à Bruxelles la mise en place de clauses miroirs vous savez pertinemment qu'elles permettent d'appliquer aux produits importés les mêmes normes de production que dans l'Union européenne, lorsque cela est pertinent et scientifiquement justifié, pour atteindre nos objectifs sanitaires et environnementaux. C'est ce que nous faisons depuis longtemps en interdisant, par exemple, l'importation de produits issus d'animaux nourris aux hormones depuis 1996 ou encore en imposant à nos partenaires de respecter les règles européennes en matière d'abattage de bovins. En janvier 2022 au plus tard, monsieur Duplomb, nous n'accepterons plus les importations dans l'Union européenne de produits issus d'animaux élevés avec des antibiotiques comme facteur de croissance pour lutter contre le phénomène mondial d'antibiorésistance.

Je voudrais également revenir sur certaines filières agricoles sensibles pour lesquelles nous faisons un suivi régulier approfondi, à savoir les viandes de boeuf, de porc et de volaille, ainsi que l'éthanol et le sucre. À l'heure actuelle, les quantités exportées depuis le Canada vers l'Union et la France sont très faibles 104 tonnes pour la viande de boeuf en France en 2019, dont seulement 45 tonnes ont profité des réductions tarifaires du CETA. C'est une goutte d'eau par rapport à la production française de 1,45 million de tonnes. Le CETA n'a donc pas eu, à ce jour, l'effet déstabilisateur que certains lui prédisaient, ... À ce jour ... ... parce qu'il ne s'oppose en rien à ce que nous appliquions nos règles d'entrée sur les marchés européens et français, qui précisent que cette viande doit avoir été nourrie sans hormones. Nous restons malgré tout vigilants : un quatrième rapport du comité de suivi est en cours de préparation et comprendra les chiffres de 2020. Il sera bien évidemment communiqué au Parlement. Sur le plan environnemental et climatique, l'étude d'impact réalisée par le Cepii en 2019 souligne clairement que l'impact du CETA sur les émissions de CO2 sera extrêmement limité, tant au niveau français qu'à l'échelle mondiale. À l'inverse, le CETA a permis d'initier des coopérations nouvelles avec nos partenaires canadiens. Nous partageons des combats communs dans le cadre du partenariat bilatéral de 2018 sur la lutte contre le changement climatique. Nous travaillons notamment sur les échanges de technologies vertes, sur la réduction des émissions du transport maritime ou encore sur la finance verte. J'entends des préoccupations concernant la protection du droit à réguler. Je vais être très clair : notre droit à réguler ne sera pas remis en cause par le CETA. le CETA. Une coopération réglementaire existe dans le cadre de cet accord, mais elle est de nature volontaire. Aucune décision modifiant le cadre réglementaire de l'Union ne peut y être adoptée : il s'agit d'une prérogative souveraine du législateur européen. Cette coopération ne peut donc en aucun cas conduire à des normes moins strictes en matière sanitaire, sociale

Ainsi, les agendas et comptes rendus des réunions sont publiés sur le site de la direction générale du commerce. En outre, la Commission consulte régulièrement les États membres, mais aussi la société civile, sur les sujets traités dans ces enceintes. Enfin, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États du CETA, qui a été évoqué voilà quelques instants, n'a plus rien à voir avec l'ancien dispositif d'arbitrage privé (ISDS), qui a suscité de nombreuses critiques légitimes.

Ce nouveau système garantit explicitement le droit à réguler des États. Le CETA reflète sur ce terrain les réformes ambitieuses portées par la France, qui s'inscrivent également dans le soutien apporté à la création sur le long terme d'une cour multilatéral d'investissements. De plus, conformément aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement et à la demande de la France, l'Union européenne et le Canada ont agréé, en janvier dernier, des textes complémentaires pour garantir le droit à réguler des États, notamment dans le domaine climatique. Ce veto climatique s'appliquera à l'ensemble de nos politiques publiques en matière non seulement climatique, mais aussi sanitaire, sociale ou culturelle, par exemple. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, notre approche en matière de politique commerciale n'est pas dogmatique, mais fondée sur des faits. Les chiffres et indicateurs montrent aujourd'hui que le CETA bénéficie à nos entreprises, à nos agriculteurs, et qu'il n'a aucun impact négatif sur le plan sanitaire ou environnemental. Je souhaite également rappeler que le Gouvernement a été proactif dès les premiers jours de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord avec la mise en place du plan d'action CETA, qui visait trois objectifs : assurer une application exemplaire de l'accord accélérer son action contre le changement climatique ; renforcer l'ambition environnementale, sanitaire, sociale de la politique commerciale européenne. Dans ce cadre, comme le Président de la République l'a rappelé, nous avons beaucoup travaillé ensemble- Gouvernement et Parlement -pour améliorer le suivi de cet accord et en évaluer mieux les effets.

Une proposition sera faite par la Commission européenne pour la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières afin de lutter contre les fuites de carbone. Le poste de procureur commercial européen en charge de la bonne application des règles en matière de commerce international et du respect des engagements pris par nos partenaires a été créé l'été dernier- il s'agit du français Denis Redonnet. la Commission a repris la demande portée par la France de faire de l'accord de Paris une clause essentielle des futurs accords commerciaux. Nous devons bien évidemment aller encore plus loin. C'est le sens du travail que nous avons réalisé avec les Pays-Bas depuis un an, ce qui a contribué à faire bouger les lignes, et de notre contribution à la revue de la politique commerciale en cours. Nous poursuivrons notre action pour une meilleure prise en compte du développement durable dans la politique européenne dans la perspective de notre présidence du Conseil de l'Union au premier semestre de 2022.

À cet égard, l'année 2021 sera particulièrement cruciale avec la tenue, en fin d'année, de la COP26. Nous attendons une ambition climatique accrue de tous les États parties à l'accord de Paris pour amplifier nos efforts de lutte contre le dérèglement climatique. Et la date

et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité, présentée par Mme Marie-Claude Varaillas, M. Gérard Lahellec et plusieurs de leurs collègues (proposition

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA, affirmait à son article 1 l'existence d'un droit à l'eau, en indiquant que « l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». En 2010, l'ONU a adopté une résolution prévoyant que « le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie ». En 2015, les États membres des Nations unies ont adopté les objectifs 2030 de développement durable, qui placent le droit humain d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène au coeur des dix-sept objectifs de développement durable. En décembre 2020, l'Union européenne a publié une directive qui vise « à améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine » et qui prévoit l'obligation pour les États membres de mettre en oeuvre le principe de l'accès à l'eau potable pour tous. Le droit à l'eau est donc clairement défini et reconnu en droit positif. aujourd'hui, ce droit demeure largement fictif, puisque aucun instrument légal ne permet de garantir concrètement son exercice et que l'accès de tous à ce service de première nécessité reste empreint de grandes inégalités tarifaires, qualitatives qualitatives et spatiales. Les faits sont têtus : selon la Fondation Abbé-Pierre, l'eau reste inabordable pour 1,2 million de personnes branchées au réseau de distribution ; plus de 140 000 personnes environ ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d'eau. Face à cette situation, les associations sont très engagées pour aller au-delà des déclarations d'intention. Il existe par ailleurs un certain nombre d'initiatives parlementaires qui ont été examinées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Malheureusement, le Sénat, à l'époque, avait totalement vidé de sa substance cette initiative. Nous remettons donc aujourd'hui l'ouvrage sur le métier. Certes, et certains de mes collègues nous l'ont rappelé en commission, il existe déjà des outils pour aider les plus fragiles à payer leur facture d'eau. La loi Brottes a ainsi permis une expérimentation de tarification sociale, qui s'applique jusqu'au 15 avril 2021- c'est aujourd'hui ! -, et l'article 15 de la loi Engagement et proximité de l'automne dernier a pérennisé dans la loi cette boîte à outils : chèque eau, allocation eau, tarification sociale et gratuité. Pour autant, le caractère optionnel de ce dispositif, en réalité assez peu utilisé par les collectivités, ne permet pas de garantir effectivement le droit à l'eau. à l'eau. Si nous considérons qu'il s'agit d'un droit universel, l'État doit adopter les mécanismes législatifs adéquats. Pour cette raison, nous proposons la mise en oeuvre d'un dispositif universel d'accès applicable en tout point du territoire et pour chacun, raccordé ou non, permettant l'égalité de tous nos concitoyens devant la loi et dans leurs droits. Pour cela, nous demandons la mise en place d'une gratuité dont le niveau est à définir. Je vous le rappelle, nous nous gardons bien de définir le niveau de gratuité, en indiquant seulement ce qui est nécessaire à la dignité humaine. Ainsi, nous estimons que nous pourrions établir cette gratuité pour tous à cinq litres par personne et par jour, ce qui représenterait un coût largement acceptable pour le service public local, quel qu'en soit le mode de gestion. Ces cinq litres correspondent à une nécessité vitale. Le coût de cette mesure serait lissé entre les usagers selon un principe de solidarité. Pour le dire clairement, le budget des collectivités n'est pas impacté, car leur participation au budget de l'eau est clairement limitée, ne pouvant aller au-delà de 2 % de l'ensemble des redevances. Leurs moyens ne sont nullement affectés par cette proposition de loi. Il s'agit donc d'un principe de solidarité au sein même des usagers. Par ailleurs, pour répondre à la nécessité de permettre l'accès à l'eau de toutes les personnes qui n'ont ni compteur ni accès, nous souhaitons la mise en place d'une obligation, à la charge des collectivités locales, de permettre l'accès à la ressource pour les plus démunis par des fontaines, sanitaires et douches publics. La plupart d'entre elles le prévoient, et la charge financière ainsi créée doit être compensée, comme le permet notre proposition de loi, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Les collectivités peuvent également solliciter

de prioriser la mise aux normes des équipements sanitaires ou des travaux sur les réseaux d'assainissement. Notons également qu'un certain nombre de collectivités s'engagent déjà dans cette voie sans attendre la loi, puisqu'il s'agit bien d'une question de respect de la dignité humaine. Je me permets de faire quatre remarques pour préciser l'opportunité politique d'adopter ce texte. Premièrement, la révision de la directive Eau de l'Union européenne nous pousse à définir des modalités d'accès pour les populations qui n'ont pas d'accès physique à l'eau. Si ce n'est fait aujourd'hui, il faudra, à l'avenir, en tenir compte. Ainsi, l'article 16 de cette directive comprend des mesures fortes telles que l'évaluation de la proportion de la population n'ayant pas accès à l'eau potable et l'encouragement à installer des fontaines gratuites dans les villes et les lieux publics, à favoriser la fourniture d'eau du robinet dans les restaurants, les cantines et les services de restauration. Il engage également les États à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à l'eau potable pour les groupes vulnérables et marginalisés. Je vous le rappelle, le droit européen s'impose. Faute de transposition, la France sera condamnée. Comment le pays des droits de l'homme peut-il assumer d'être en retard sur un tel sujet ? Deuxièmement, la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à repenser la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement, pour des questions de santé et de salubrité. Les gestes barrières nécessitent l'accès à l'eau. Le « quoi qu'il en coûte » doit, dans ce domaine aussi, prévaloir. Le Gouvernement a ainsi pris, le 27 mars 2020, des dispositions pour que les préfets et les collectivités locales assument leurs responsabilités en la matière notamment à ce que soit garanti l'accès à l'eau, à des sanitaires, à des douches et à des laveries. Cela doit perdurer. La sixième puissance mondiale doit pouvoir financer les équipements nécessaires à la dignité de nos concitoyens. risque de gaspillage de la ressource n'est pas justifié, alors que la consommation moyenne constatée est de cent quarante litres par jour et par personne. Comme le préconisent les associations pour la défense du droit à l'eau, il pourrait s'agir de la mise à disposition de cinq litres gratuits

La compétence « eau et assainissement » n'est pas retirée aux collectivités ; la liberté de l'organiser selon leur choix non plus. La gratuité que nous proposons est donc un socle qui n'empêche nullement les collectivités en question de compléter ce dispositif par l'un des outils de l'article 15 de loi Engagement et proximité.

le Conseil constitutionnel a déjà jugé, notamment pour ce qui concerne la loi SRU, qui impose aux collectivités la construction de logements sociaux, qu'une telle contrainte était acceptable. Ainsi, les conditions d'intervention du législateur ont été précisées dans la décision du 7 décembre 2000. été indiqué que les obligations et les charges auxquelles la loi assujettit les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent répondre à « des exigences constitutionnelles » ou concourir à « des fins d'intérêt général ». Nous pouvons tous le comprendre, la fin d'intérêt général de garantir à tous l'accès à l'eau justifie dans des proportions raisonnables l'intervention du législateur. Sur le fond, le fond, nous voulons opposer le modèle de la gratuité et, donc, de la solidarité à celui de la marchandisation, non pas de manière dogmatique, mais en instaurant une part de gratuité, quitte à l'élargir par la suite. Sans aller jusqu'à faire du droit à l'eau un droit opposable à l'image du droit au logement opposable, le DALO, il convient de définir un cadre légal pour donner corps et et contenu à ce droit défini comme un droit fondamental par l'ONU. Il convient donc pour partie de s'extraire de la notion d'« aide aux ménages », dont la dimension caritative est trop réductrice, pour s'orienter vers celle d'un droit directement applicable à l'ensemble de nos concitoyens et, donc, universel. C'est dans ce cadre que la notion et l'outil de la gratuité sont des leviers puissants, à la fois d'égalité sociale et territoriale, ainsi que d'universalité. En effet, cela place le débat non pas sur le terrain de l'accompagnement social de personnes en difficulté, mais bien sur celui de l'affirmation d'un droit de portée générale et universelle, conformément à l'esprit de la LEMA et des engagements internationaux de la France. La parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en préambule, je souhaite rappeler la conviction qui a animé et guidé mon travail de rapporteur.

Au terme des auditions que j'ai menées, il m'est apparu avec la force de l'évidence que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit vital, dont dépendent la survie, mais aussi la santé, l'hygiène et la dignité de toute femme et de tout homme. Des publications scientifiques ont nourri le débat public de données alarmantes et de chiffres vertigineux. Il y a là un sujet dont personne ne peut se désintéresser, qui s'aggrave et m'apparaît à certains égards comme le « défi du siècle ». La relative abondance de l'eau en France nous empêche parfois de percevoir l'urgence d'agir et les effets de l'exclusion de l'eau. Nous considérons un robinet ou une fontaine comme un élément banal qui ne retient plus l'attention. En effet, loin est le temps où l'eau était à aller chercher plus qu'elle ne venait pas à nous. Figurez-vous que je suis né à quatre kilomètres du bourg de Plufur, un petit village des Côtes-d'Armor. Quand j'étais petit, mes petits camarades qui habitaient au bourg allaient jusqu'au robinet du village pour pouvoir avoir de l'eau.

vite. Ces robinets n'en constituaient pas moins un véritable service public de l'eau, auquel chacun avait accès ... plus ou moins rapidement. N'oublions pas que si, aujourd'hui, nous sommes nombreux à bénéficier de l'eau courante, obtenue sans courir,

Avec l'air, l'eau est en effet la ressource vitale, essentielle à la vie et aux activités économiques. Sans un accès sécurisé à une eau potable de bonne qualité, l'être humain reste tributaire de la satisfaction de ce besoin : pas de dignité possible, pas de développement durable, pas de justice sociale, pas d'accès aux fruits de la croissance ! Je suis convaincu qu'il ne se trouve personne dans cet hémicycle pour s'opposer à l'idée que l'eau potable est un bien commun dont aucun être humain ne devrait être exclu. C'est aussi ce que j'ai perçu au sein de la commission lors de nos débats.

Le droit à l'eau progresse ; il se constitutionnalise dans certains pays ; il est reconnu par l'Organisation des Nations unies. Des pays et des collectivités ont d'ores et déjà instauré la gratuité des premiers volumes. La prise de conscience existe également au niveau européen la nouvelle directive européenne sur l'eau potable, de décembre 2020, en constitue un parfait exemple. Nous n'arrivons donc pas sur un terrain vierge de toute avancée. Je ne vous demande pas d'être révolutionnaires ni d'aller à l'encontre de vos sensibilités politiques il s'agit simplement de parfaire l'oeuvre déjà accomplie, dans un esprit humaniste. Ce droit est reconnu, proclamé et consacré. Mais il y a le droit et il y a le fait. Or le droit, insuffisamment opposable et trop souvent déclaratoire, ne reflète pas le fait. Aujourd'hui, 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas un accès sécurisé à l'eau potable. potable. Notre pays n'est pas épargné par certaines formes de précarité en eau. Il y a les « exclus de l'eau » : 1,4 million de Français métropolitains, les personnes sans domicile fixe ou vivant dans des habitats de fortune. Il existe aussi les « précaires en eau les ménages consacrant plus de 3 % de leur budget à payer leurs factures d'eau. Ils représentent, selon les associations que j'ai entendues, plus de 1 million de personnes. Voilà pour ce qui est de l'écart entre le droit et le fait. Le législateur n'est pas resté insensible à cette question et a essayé, compte tenu de l'écart existant, de rendre le droit plus effectif. La loi Brottes de 2013 a interdit les coupures d'eau des ménages pour impayés et a mis en oeuvre une expérimentation de tarification sociale de l'eau. À la différence des aides curatives, ponctuelles, partielles et non automatiques, les aides préventives s'appliquent dès lors que le foyer satisfait aux critères prédéfinis et prennent la forme soit d'une tarification intégrant une première tranche dite sociale

Face à ce constat, il est nécessaire de consolider les acquis en garantissant de manière encore plus effective le droit d'accès à l'eau. L'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût, qui est celui de son acheminement, de son traitement et de son assainissement. Les services de l'eau, industriels et commerciaux, reposent sur une logique de tarification à l'usager bénéficiaire, et non sur un financement par l'impôt. En vertu de la libre administration des collectivités territoriales, les communes et EPCI qui en assurent la distribution sont libres de mettre en oeuvre des politiques locales en vue de favoriser l'accès de l'eau aux populations précaires ou marginalisées.

Il instaure uniquement la gratuité d'une volumétrie essentielle, indispensable à la vie et à la dignité. Le surplus, au-delà ce qui est nécessaire pour étancher sa soif et pourvoir à son hygiène, continuerait bien entendu à faire l'objet d'une facturation à l'usager, pour ne pas remettre en cause l'équilibre financier des collectivités gestionnaires ou délégantes. J'achèverai mon propos en citant la directive européenne sur l'eau potable, qui enjoint aux États européens l'installation d'« équipements dans les espaces publics, lorsque cela est techniquement réalisable Le texte que nous examinons aujourd'hui est l'occasion d'en commencer la transposition et de garantir véritablement un droit à l'eau pour tous en France. Le bloc communal serait responsable de la mise en oeuvre de cette noble mission, au plus près des besoins, en vertu du principe constitutionnel de subsidiarité. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas adopté cette proposition de loi. À titre personnel, vous l'aurez compris, j'y suis toutefois favorable.

mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui est soumise à votre examen vise à garantir le droit à l'eau par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d'eau potable et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité. En France, l'eau est un bien commun de la Nation et son usage appartient à tous. Notre droit consacre d'ores et déjà cet objectif. Le code de l'environnement établit que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables L'accès à l'eau pour tous est évidemment un objectif que je partage et auquel le Gouvernement souscrit pleinement. À cet égard, les articles 19 et 19 du projet de loi Climat et résilience,

en rassurant très vite les Français sur la qualité et la sécurité de l'eau du robinet. Toutefois, aujourd'hui encore, en 2021, 235 000 personnes sont privées d'un accès permanent à l'eau. Ce n'est pas acceptable, et nul ne peut s'y résoudre. Nous avons encore du travail pour assurer à chacun l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est pour répondre à cet objectif que le Gouvernement a lancé la réforme de la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe.

Il veillera à la continuité du service et réalisera tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux. Il était temps de répondre à ce besoin essentiel, que nous nous devons d'assurer à tous les Guadeloupéens. Dans le même temps, le Gouvernement mobilise 300 millions d'euros du plan France Relance, pour sécuriser et moderniser les infrastructures de distribution d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Les agences de l'eau et l'OFB en assurent le pilotage. Ces crédits sont déjà largement engagés, ce qui montre bien la mobilisation des collectivités sur cette mission fondamentale. Si la ressource en eau est un bien public inaliénable, l'accès à ce bien repose sur un service rendu, qui a un coût. En France, le prix de l'eau qui est facturé à l'usager correspond au prix du service comprenant le prélèvement, le traitement, la distribution et les réseaux. distribution et les réseaux. Il est fixé localement par la collectivité- la commune ou l'intercommunalité -ou par le syndicat d'eau potable auquel elle a confié l'organisation du service. Les collectivités organisatrices peuvent choisir d'exploiter directement le service dont elles ont la responsabilité en régie ou d'en déléguer l'exploitation

d'eau. Dans le cadre de la loi Brottes de 2013, qui a interdit la pratique des coupures d'eau pour une résidence principale, même en cas d'impayés, une expérimentation a été menée auprès de cinquante collectivités en vue de tester différentes politiques sociales en faveur de l'accès à l'eau. Cette expérimentation a montré l'importance du principe de subsidiarité. En fonction de ses caractéristiques et des enjeux qui lui sont propres, chaque collectivité participante a pu mettre en place des mesures spécifiques et adaptées à son territoire et à son organisation. En raison de ce succès, les mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ont été élargies à l'ensemble des collectivités et pérennisées dans la loi Engagement et proximité de 2019. Les collectivités sont donc déjà en mesure de mettre en place des dispositifs qui font l'objet de la présente présente proposition de loi, comme la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'aides au paiement des factures, ou encore des mesures favorisant les économies d'eau. La possibilité de rendre les premiers mètres cubes gratuits existe déjà, mais, on le sait, cette gratuité est à observer avec précaution, car elle peut avoir un effet contraire à nos objectifs de bonne gestion de la ressource et de maîtrise des consommations.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'eau est un enjeu pour de nombreuses régions du monde, y compris en France. Les situations de stress hydrique sont de plus en plus fréquentes et provoquent des tensions. Cela a un impact sur les populations et sur de nombreux territoires. Si l'eau recouvre une surface importante de notre planète et travaille à son équilibre, elle est surtout une part cruciale du corps humain. N'oublions jamais que nous sommes nous-mêmes constitués à 60 % d'eau. L'accès à l'eau et sa qualité sont donc indispensables à la vie. Cette proposition de loi, dont nous saluons l'esprit, évoque dans l'exposé des motifs l'objectif n° 6 de développement durable proposé par les Nations unies, consacré à l'eau et à l'assainissement. Encore un tiers de l'humanité n'a pas accès à un assainissement convenable en matière d'eau, et la gestion durable de cette ressource n'est pour le moment pas assurée comme il le faudrait dans de nombreuses parties du monde. En France, nous avons la chance d'avoir accès à une eau de bonne qualité au robinet grâce à des réseaux et des systèmes d'assainissement efficaces. Cependant, environ 1 % de la population n'est pas raccordée à un approvisionnement public en eau potable. Ce n'est pas acceptable. Nous connaissons les sujets tels que le vieillissement des infrastructures dans certains de nos territoires, ou encore l'adaptation des réseaux à de nouveaux enjeux comme le changement climatique. Le directeur général de Suez rappelait il y a quelques jours que l'investissement dans l'eau et l'assainissement s'élevait à hauteur de 6,5 milliards d'euros par an. Il a même ajouté que les besoins allaient nécessiter une multiplication par deux des investissements. Une nouvelle fois, la crise que nous traversons a mis en exergue le caractère indispensable de l'hygiène et de l'accessibilité à l'eau potable. L'accès à l'eau et sa constante amélioration, notamment pour les personnes les plus vulnérables, sont des objectifs à atteindre sur l'ensemble du territoire. Le Sénat travaille de manière régulière sur le sujet. Les discussions autour du texte en commission ont fait ressortir ce point. Encore récemment, lors de l'adoption de la loi Engagement et proximité, le système de tarification sociale de l'eau a été renforcé et étendu. Ainsi, il existe déjà des possibilités pour les collectivités territoriales de moduler les tarifs pour permettre un accès à l'eau et à l'assainissement pour le plus grand nombre. Nos élus locaux, fins connaisseurs de leurs territoires, endossent des responsabilités importantes sur ce sujet. La gratuité des premiers volumes d'eau, qui est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi, fait partie des possibilités offertes aux territoires dans la gestion du prix de l'eau. Il est important sur ce sujet que les collectivités puissent mettre en place les outils qui sont le plus appropriés en fonction des besoins de leur population et des contraintes auxquelles elles doivent faire face. Comme cela a déjà été souligné, les dispositions imaginées dans cette proposition de loi ne semblent pas répondre à la flexibilité requise ni aux avancées qui ont déjà eu lieu au niveau local. Nous soutenons l'objectif d'un accès pour tous à l'eau potable de qualité, mais nous pensons que des outils existent et qu'il faut d'abord une bonne application des règles en vigueur. Il convient de laisser le temps et l'espace aux collectivités d'utiliser et de mettre en place les possibilités qui leur sont données afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous pour tous nos concitoyens, en fonction des spécificités locales. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants s'abstiendra sur cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'accès à l'eau est un droit fondamental et élémentaire. L'eau est un bien commun qui ne peut être accaparé et dont l'accès doit être garanti à chacun et chacune. La question du droit à l'accès à l'eau pour toutes et tous est donc un enjeu essentiel, et nous souhaitons rappeler, avec le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, combien cette question mêle étroitement à la question écologique de préservation des ressources les enjeux de justice sociale et de santé publique. L'eau est un patrimoine commun, mais aussi un patrimoine partagé, qui vient à manquer. Elle est également une ressource précieuse qu'il faut protéger. Seulement 44 % des eaux de surface étaient évaluées en bon ou très bon état en 2015. La préservation et l'accès aux ressources en eau potable sont des questions écologiques cruciales, à l'heure où le dérèglement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles représentent un obstacle en plus qui privera les populations les plus vulnérables de cette ressource. Dans le monde, ce sont près de 2,2 milliards de personnes qui sont encore privées d'accès à l'eau, et plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr. La France n'échappe pas à cette problématique grave. On estime à environ 300 000 le nombre de personnes privées d'un accès à un réseau d'eau, à des toilettes et à des douches. Un million de ménages précaires sont dans la difficulté pour payer leur facture d'eau. Alors, où est le droit fondamental de l'accès à l'eau potable et à une hygiène de qualité ? Comment garantir un besoin aussi vital pour chacune et chacun ? C'est bien l'objet de cette proposition de loi que de combler cette inégalité,

Dix ans après l'ONU, qui proclamait que l'eau est un droit humain fondamental, l'Union européenne, en décembre 2020, a publié une directive qui vise à « améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine » et qui contient l'obligation pour les États membres de mettre en oeuvre le principe de l'eau potable pour tous. La directive dispose ainsi que « les États prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés ». Des mesures à la hauteur des ambitions de la directive doivent être prises dans le cadre de sa transposition. Cette proposition de loi pourrait en constituer un très bon commencement. La directive devra tôt ou tard être transposée en droit français. Alors, saisissons l'opportunité et permettons au Parlement de se positionner sur le texte et d'en dessiner les contours. Prévoir dans le code de la santé publique que chacun doit Prévoir dans le code de la santé publique que chacun doit avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement, prévoir aussi la mise à disposition gratuite d'équipements au plus près des populations : autant de premiers pas vers la garantie concrète de ce droit. droit. Une aide préventive pour les ménages, afin que la facture d'eau ne dépasse pas 3 % de leurs ressources, est aussi de nature à répondre à l'esprit et aux objectifs de la directive. En effet, même si l'on salue les dispositifs sociaux mis en place en droit français ces dernières années, on ne peut que déplorer le fait que les aides soient conditionnées à l'existence de compteurs individuels et que le montant moyen des allocations reste dérisoire. Par ailleurs, des craintes ont été exprimées sur les nouvelles charges que la gratuité des premiers mètres cubes et la mise à disposition des équipements pourraient induire pour les collectivités. Cependant, la mise en place de la gratuité va permettre de diminuer le nombre d'impayés d'eau et, donc, de décharger les centres communaux d'action sociale et les fonds de solidarité pour le logement. Les collectivités pourraient mettre à disposition les équipements sanitaires et de distribution d'eau dans des bâtiments publics ou appartenant à des associations subventionnées. Ils pourraient aussi être financés par une tarification sociale progressive de l'eau. Le droit fondamental d'accès à l'eau doit être garanti pour toutes et tous, car il s'agit de la satisfaction de besoins élémentaires nécessaires à la bonne santé publique. Thomas Sankara disait : « Il faut choisir

Pour garantir que chaque individu ait accès à ce bien commun de l'humanité, et au vu des enjeux renforcés par l'urgence écologique, il est nécessaire d'avancer contre l'accaparement des ressources en eau par des intérêts privés dans une logique de profit,

par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d'eau potable et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité. Ce texte est discuté quelques semaines après la journée mondiale de l'eau, un événement qui nous a rappelé l'importance du défi que représente la préservation de ce bien essentiel et fondamental pour les années à venir. L'eau, c'est la vie, les enjeux sont considérables. Les dommages environnementaux, associés aux changements climatiques, sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde. Les inondations, la sécheresse et la pollution sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs. L'objectif de développement durable n° 6 a été adopté par les États membres des Nations unies à l'horizon de 2030. Il a notamment pour cible de réduire de moitié la proportion d'eaux usées non traitées et d'augmenter considérablement le recyclage et la réutilisation. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est reconnu comme un droit de l'homme depuis 2010. Pourtant, près de 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès aujourd'hui à des services d'alimentation domestique en eau potable gérés en toute sécurité et près de 2,6 millions meurent chaque année de maladies liées à l'eau, l'une des premières causes de mortalité au monde. L'accès à l'eau et à l'assainissement est un enjeu social, environnemental, mais aussi économique. En France, depuis quinze ans, le cadre juridique a évolué. Il permet aux collectivités locales et à leurs établissements publics d'adapter leurs politiques tarifaires. L'article 1 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 dispose que « l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». En 2013, la loi la loi Brottes a ouvert la possibilité pour les collectivités locales de mettre en oeuvre l'expérimentation pour une tarification sociale de l'eau. Cette loi a d'ailleurs montré l'importance du principe de subsidiarité dans ce domaine. La loi Engagement et proximité de 2019 a quant à elle introduit pour toutes les collectivités la possibilité de mettre en place les mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau de leur choix. Toutes les collectivités ont donc déjà la faculté de mettre en place un éventail de mesures sans souffrir de l'ingérence de l'État. Pourtant, selon l'OMS, en 2019, 1,4 million de Français n'avaient pas d'accès à une eau « sanitairement sécurisée 1 million de nos concitoyens consacraient plus de 3 % de leur budget mensuel à l'eau et 235 000 personnes étaient des « exclus de l'eau ». Sur ce point, la directive européenne sur l'eau potable de décembre 2020 dispose que les États européens devront se doter « d'équipements intérieurs et extérieurs dans les espaces publics, [ ...] d'une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques ». J'appelle de mes voeux une transposition rapide de cette Nous connaissons ici les réalités de la gestion locale. Si l'eau n'a pas de prix, elle a un coût ... La loi NOTRe a accéléré les transferts des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI. Quels en sont les premiers enseignements ? Un litre sur cinq d'eau traitée et mise en distribution en France est perdu. C'est l'équivalent de la consommation de 18,5 millions d'habitants. En cause, un sous-investissement important dans des réseaux de distribution vieillissants. Les transferts ont permis de disposer d'une meilleure connaissance des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif. Au rythme actuel des investissements, le renouvellement théorique s'établit à plus de cent cinquante ans, pour un budget annuel de 1,5 milliard d'euros. C'est insuffisant Concrètement, la gestion passera par des moyens supplémentaires en gestion patrimoniale, en recherche de fuites, en réparation et renouvellement des conduites, ce qui affectera le prix de ces services. Avec le réchauffement climatique, plusieurs territoires sont exposés à des phénomènes de stress hydrique : l'eau est rare. L'accès gratuit aux premiers mètres cubes d'eau et à l'assainissement est un exercice difficile. les collectivités locales et leurs établissements ont toute latitude pour mettre en place une tarification différenciée, en proposant notamment les premiers mètres cubes, qu'on appelle souvent « l'eau vitale », à des tarifs très bas. Pour y avoir travaillé sur ma communauté de communes du Pays des Abers, je vous assure que l'exercice tient de la quadrature du cercle. La compétence y est exercée en régie directe depuis 2018, pour un territoire d'un peu plus de 40 000 habitants. Nous avons Nous avons mis en place une tarification très faible sur les premiers mètres cubes et des tarifs progressifs sur les mètres cubes suivants. Plus on consomme, plus le mètre cube coûte cher. Comment concilier tarification sociale, équilibre économique et préservation de la ressource ? Toucher à l'un des paramètres provoque un déséquilibre global. L'alimentation en eau potable et l'assainissement sont des compétences des collectivités territoriales, qu'elles gèrent selon le principe de libre administration. Faisons leur confiance et laissons-les gérer leurs services en fonction des réalités de leurs territoires. Il ne peut y avoir de réponse unique et centralisée à tant de situations particulières.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le droit d'accéder à l'eau potable est inscrit dans la résolution de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 28 juillet 2010 comme un droit fondamental « essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme ». ». Chaque être humain a droit à un approvisionnement en eau potable suffisant pour vivre dans la dignité, à un coût abordable pour les usages personnels et domestiques. un nouvel article dans le code de la santé publique, selon lequel les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale prennent les mesures pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d'un raccordement au réseau. Ces collectivités sont également tenues d'installer et d'entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable, des douches gratuites pour celles de plus de 15 000 habitants, ou encore des toilettes publiques gratuites pour les communes de plus de 3 500 habitants. Le droit à l'eau est déjà inscrit dans notre droit positif, à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. La loi Brottes, en 2013, a interdit les coupures d'eau pour les résidences principales en cas de non-paiement des factures, ou encore la réduction du débit d'eau. au quotidien, force est de constater qu'il y a un fossé entre les principes et la réalité, et près de 1 million de Français rencontrent des difficultés à payer leur facture d'eau. Dans le passé, plusieurs propositions de loi ont tenté, sans succès, de garantir ce droit à l'eau. Celle que nous examinons prévoit la gratuité des premiers mètres cubes et me replonge plusieurs années en arrière.

j'ai dû me résoudre à appliquer une tarification à la consommation dès les premiers mètres cubes, mais également à augmenter le prix de l'eau, car on m'a imposé l'équilibre financier du service. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup progressé à force de politiques de gribouille dans ce domaine, un pas en avant, deux pas en arrière. De très fortes inégalités territoriales persistent, quel que soit le mode de gestion choisi- en régie municipale ou par une société privée en délégation de service public et 235 000 Français sont privés d'un accès permanent à l'eau. Une étude sur le prix de l'eau, publiée en 2018 par UFC-Que Choisir, a passé au crible 1 000 factures de collectivités territoriales représentatives, y compris en zone rurale. Elle révèle des écarts énormes, traduisant parfois des réalités géographiques, mais aussi des dérives en matière de gouvernance de la gestion de l'eau. Cette question est préoccupante, même si de nombreux services de l'eau sont exemplaires. Les Français ne sont pas égaux face au prix du mètre cube d'eau, qui varie entre 2,68 et 8,46 euros. Ce grand écart frappe aussi la région Sud-Ouest, où la fourchette va de 2,94 à 7,07 euros. le prix du mètre cube peut atteindre celui d'une bouteille de vin ! Ce prix du mètre cube n'est pas le seul facteur à prendre en compte. L'accès à l'eau comporte des coûts d'abonnement, de remboursement d'emprunts, de location de compteur ou encore de télérelevé. Ce service est aujourd'hui défini comme un service public industriel et commercial,

pour tous, et non comme un service industriel et commercial. Il n'empêche qu'il n'y a pas d'eau gratuite, quel que soit le mode de distribution choisi. La proposition de loi prévoit d'ailleurs, à son article 4, de compenser ce coût. Si l'usager ne paie pas, c'est le contribuable qui devra payer, à moins de mettre des bassines sur les terrasses et dans les jardins pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons besoin de rationaliser la gouvernance du secteur et de choisir clairement une politique sociale de l'eau

le texte que nous examinons se propose de rendre effectif le « droit à l'eau » par la mise en oeuvre de deux mesures concrètes : premièrement, l'installation dans l'espace public par les communes et les EPCI compétents de fontaines, douches et sanitaires à disposition du public deuxièmement, l'instauration de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau consommés par les ménages. Le but visé par ce présent texte est tout à fait légitime : l'accès à l'eau, et à une eau de qualité, nécessaire à l'hydratation et à l'hygiène, doit en effet être considéré comme primordial. Il en va de même du droit à l'assainissement. Ce droit a été reconnu par plusieurs textes de droit international et européen. Récemment encore, une directive européenne du 16 décembre 2020 a affirmé le droit de tous à l'eau potable, fixé de nouvelles exigences de qualité et prévu également des mesures d'information du public sur l'eau qu'il consomme. l'eau qu'il consomme. En France, le législateur a consacré dans la loi du 30 décembre 2006 « le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous Pour rendre ce droit effectif, des mesures destinées aux ménages ayant du mal à régler leurs factures d'eau ont été mises en place. Premièrement, la loi du 7 février 2011 permet aux collectivités et EPCI compétents de verser des subventions au Fonds de solidarité pour le logement afin de financer des aides versées en cas de cumul d'impayés. Par ailleurs, les impayés ne donnent plus lieu à une coupure d'eau, comme cela était le cas auparavant. Deuxièmement, le législateur a introduit en 2013 la possibilité pour des collectivités de mettre en place une tarification sociale de l'eau à titre expérimental. Enfin, la loi Engagement et proximité de 2019 a élargi cette faculté à l'ensemble des collectivités. La tarification sociale inscrite par le législateur dans le code général des collectivités territoriales- -offre beaucoup de latitude aux conseils municipaux et communautaires en ce qui concerne les modalités d'application. Les élus locaux peuvent choisir entre des tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou encore une aide à l'accès à l'eau. On constate que l'instauration d'une aide préventive réclamée par le présent texte est déjà possible pour les collectivités qui le souhaitent. Par exception, la tarification sociale peut-être financée sur le budget général, à condition de ne pas dépasser 2 % du budget spécialisé « eau ». Une proposition de loi semblable dans ses objectifs à celle que nous examinons aujourd'hui avait été votée par les députés en 2016, mais elle n'avait pas convaincu les sénateurs. Hélas, à l'instar de la proposition de loi de 2016, le texte que nous examinons présente à notre avis d'importants défauts. En ce qui concerne la gratuité de l'eau potable nécessaire aux besoins élémentaires prévue par l'article 1, plusieurs questions se posent. Premièrement, quelle serait l'articulation de cette gratuité avec la tarification sociale inscrite dans la loi et déjà mise en place dans de nombreuses communes ? La présente proposition de loi ne mentionne ni ces aides existantes ni leur articulation avec la gratuité qu'elle prévoit d'instaurer. La superposition de ces deux dispositifs d'aide ne nous paraît ni d'une grande efficacité ni d'une grande lisibilité pour nos concitoyens. Deuxièmement, se pose la question du financement. L'eau et l'assainissement doivent faire l'objet de budgets annexes, « étanches »- si j'ose dire -par rapport au budget général des collectivités et de leurs EPCI, sauf exception, comme celle qui est prévue par la loi Engagement et proximité que j'ai évoquée. L'absence d'étude d'impact ainsi que l'imprécision quant à la quantité d'eau concernée ne permettent pas d'avoir une idée précise du manque à gagner que les gestionnaires de service public d'eau devront combler. De plus, la dotation globale de fonctionnement ne peut abonder ces budgets « eau » et « assainissement ». Dès lors, quoi qu'en dise l'article 4 du présent texte, il ne fait guère de doute que la gratuité instaurée créera un manque à gagner que les collectivités gestionnaires devront compenser

Le financement de ces installations repose sur les municipalités et les EPCI compétents. Je déplore l'absence d'information, tant sur le nombre actuel de ces installations dans les communes concernées que sur les besoins estimés des populations pour ce genre d'infrastructures. Il est ainsi difficile d'évaluer l'effort financier à réaliser. Au fond, ne serait-il pas préférable de faire confiance à l'échelon local pour satisfaire les besoins de sa population en eau dans l'espace public ? Dans la commune de 1 000 habitants dont j'ai eu l'honneur d'être maire, nous avons déjà des toilettes publiques gratuites et accessibles aux handicapés. Je connais de nombreuses communes d'une taille inférieure au seuil retenu par la présente proposition de loi qui ont fait de même sans qu'il soit besoin de légiférer. Comme l'avait fait le groupe Union Centriste lors de l'examen du présent texte en 2017, je déplore que les outre-mer, où la question de l'eau et de l'assainissement est si différente de la métropole, ne bénéficient pas d'un régime adapté à leurs spécificités dans le présent texte. Autre regret : l'absence de mesures d'information et de sensibilisation à destination du public, notamment des plus jeunes, autour de l'eau et de l'assainissement. l'assainissement. Mes chers collègues, du fait des raisons que j'ai évoquées précédemment, le groupe Union Centriste ne votera pas ce texte. Nous estimons que la législation actuelle assure en grande partie l'effectivité du droit à l'eau de l'ensemble de nos concitoyens et présente de plus l'avantage de laisser aux élus locaux une liberté de choix bienvenue quant aux modalités d'application de la tarification sociale de l'eau. sans doute être envisagées. Il faudrait en premier lieu pouvoir dénombrer mieux que ce n'est le cas aujourd'hui celles et ceux qui ont des difficultés à accéder à l'eau potable et connaître avec plus de précision leurs besoins en eau, tant dans l'espace public que privé. que l'ajout d'un mécanisme préventif supplémentaire, incertain quant à ses conséquences, particulièrement rigide et uniforme dans son application, et qui conduirait inéluctablement à créer un manque à gagner pour les collectivités gestionnaires, ne nous semble pas souhaitable. La parole

je remercie Marie-Claude Varaillas et les membres du groupe CRCE de cette proposition de loi, qui nous permet de porter à nouveau dans l'hémicycle la question du droit à l'eau, un droit essentiel quant à l'évolution duquel nous restons, en France, bien timides. Le droit à l'eau pour tous : posons enfin ce principe universel ! Le texte que nous examinons affirme un droit à l'eau potable et à l'assainissement pour chacun, c'est-à-dire le droit de disposer d'une quantité d'eau qui, chaque jour, permette de répondre aux besoins élémentaires et d'accéder à des équipements pour assurer le minimum d'hygiène et de dignité d'un être humain. c'est bien de notre humanité qu'il est question et d'un bien collectif, d'un bien commun indispensable à la vie. Ce texte prévoit également l'obligation, pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'assurer l'installation et l'entretien d'équipements permettant la distribution d'eau potable, ainsi que de toilettes et de douches publiques d'accès gratuit en fonction de certains seuils démographiques. Il fixe enfin la gratuité d'un volume d'eau potable minimum pour l'alimentation et l'hygiène de chaque individu.

depuis 1992, la loi reconnaît la ressource en eau comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation. La loi Brottes du 15 avril 2013 a permis l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau pour cinq ans, ouvrant la voie à la définition de tarifs adaptés aux difficultés de certains foyers. l'attribution d'aides au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau. En avril 2018, nos collègues Monique Lubin et Éric Kerrouche déposaient une proposition de loi visant à proroger cette expérimentation. Nous constatons toutefois que peu de syndicats des eaux ont totalement mis en oeuvre le dispositif. Le système de prise en charge de ces besoins en eau pour les individus et les familles en situation de précarité reste complexe et montre ses limites. Envisager la gratuité de la ressource en eau encadrée par la loi est donc une solution qui pourrait se révéler moins onéreuse que le coût du traitement social actuel. Je vous invite à y réfléchir, mes chers collègues. Malgré ces dispositions législatives, auxquelles s'ajoute l'interdiction des coupures d'eau et de réduction du débit, le droit à l'eau n'est pas effectivement garanti et ne parvient pas à être consacré pleinement dans notre pays. C'est pourtant avec le soutien de la France qu'il y a plus de dix ans, en juillet 2010, l'assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution reconnaissant le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Certains pays, comme l'Uruguay et la Slovénie, l'ont déjà introduit dans leur Constitution. Depuis, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur en termes de santé, de développement et d'environnement. N'oublions pas que ce droit compte parmi les dix-sept objectifs 2030 de développement durable adoptés par les États membres des Nations unies. De nombreuses associations, organisations humanitaires, caritatives et environnementales nous interpellent depuis de nombreuses années. La fondation France Libertés et la Coalition Eau en sont les fers de lance. Dans le monde, 2,2 milliards d'êtres humains ne disposent pas d'accès sécurisé à l'eau potable et 4,2 milliards à l'assainissement. Plus de 2,6 millions de personnes, dont une majorité d'enfants en bas âge, meurent chaque année de maladies liées à la consommation d'une eau impropre.

1 million de familles ne sont pas en capacité de régler leur facture d'eau. Nous ne pouvons ignorer ces chiffres. L'accès à l'eau pour des populations déjà fragilisées et souvent fortement marginalisées est vital, humainement mais aussi socialement. Quelle insertion sociale, scolaire et professionnelle est possible pour ces personnes si ce droit fondamental n'est pas respecté par notre République ? C'est une simple question de dignité et d'égalité. La crise sanitaire actuelle met en lumière l'importance vitale de l'hygiène pour prévenir et endiguer les maladies. Les autorités recommandent de manière répétée de se laver les mains. Comment répondre à cette exigence quand on est privé d'accès à l'eau ? Garantir à tous un droit à l'eau dans ce contexte, n'est-ce pas aussi nous protéger tous ? Ceux qui s'opposent à la gratuité de l'eau, vitale et enjeu de santé publique, s'opposeraient-ils aussi à la gratuité des vaccins ? La covid-19 a bousculé nos habitudes, nos schémas de gestion des finances publiques et des ressources pour envisager une solidarité, un partage comme cela ne s'était pas produit dans notre pays depuis plusieurs décennies. L'eau en partage, l'eau accessible à tous, doit être posée comme un principe fondateur et indiscutable de notre vivre ensemble. C'est une ressource vitale, à présent cotée en bourse, sans cesse menacée de financiarisation et objet de spéculations sur un marché qui nie la priorité des besoins humains et ignore la valeur de l'eau pour en fixer le prix un paradoxe dangereux. « L'eau pour la vie, pas pour le profit », affirmait une tribune publiée dans par 550 organisations et collectifs de la société civile à l'occasion de la journée mondiale de l'eau organisée le 22 mars dernier. Les enjeux sont majeurs, comme l'illustre le récent et titanesque affrontement Suez-Veolia. Dans la perspective plus globale du réchauffement climatique et des enjeux de développement durable, défendre le principe d'un droit à l'eau est incontournable. Laisserons-nous au marché la gestion et la répartition de l'eau ? Protégeons donc ce bien commun ! Les solutions existent. Affirmer le droit à l'eau potable et à l'assainissement et assurer la mise à disposition d'équipements sanitaires et de distribution d'eau répond aux besoins essentiels d'une population que l'on peut dénombrer. Sur ce fondement, nous le savons, la dépense est acceptable. Contenue et encadrée, elle ne fragiliserait pas les équilibres de gestion de nos collectivités, qu'il faut accompagner. Il serait envisageable de rendre ce dispositif plus lisible et de permettre aux gestionnaires de l'intégrer dans leur modèle économique, en inscrivant dans la loi ce volume d'eau gratuit afin d'en limiter le coût potentiel et d'agir en respect des règles de recevabilité financière existantes.

donc prévoir. La répartition du surcoût se fera à partir de seize mètres cubes et au-delà. Les plus précaires, moins consommateurs, bénéficieraient ainsi de la gratuité de l'eau qui leur est indispensable, tandis que les foyers plus favorisés et aussi plus consommateurs assumeraient collectivement et de façon raisonnablement répartie le coût de cette solidarité. Plus on consomme, plus on paye : dans le contexte actuel, J'ajoute que les gains d'efficacité des réseaux pour éviter les pertes permettraient largement de compenser la gratuité des premiers mètres cubes. Non, la gratuité n'ouvre pas nécessairement la voie aux abus et à l'augmentation de la consommation. La gratuité des premiers mètres cubes ne menace en aucun cas les compétences des collectivités territoriales en matière d'assainissement collectif et non collectif et n'ouvre pas la voie à la multiplication des installations illégales. Il faut faire confiance à la population, mais aussi aux collectivités pour instaurer et gérer cet accès à l'eau tout en leur en donnant les moyens. Les accompagner constituerait sans aucun doute un acte politique fort, affirmant le droit à l'eau pour tous, principe de portée universelle lié aux droits humains. Si nous en avons la volonté, ce principe encadré deviendra un outil précieux pour nos élus locaux confrontés à des situations parfois inextricables aux plans humain et sanitaire face à ceux qui sont privés d'eau. Peut-on accepter que la France, sixième puissance mondiale en 2021, refuse ce droit essentiel aux plus précaires sur le territoire des droits de l'homme ? Il est temps de traduire dans la loi les engagements nationaux et internationaux de notre pays pour le respect des droits fondamentaux de la dignité humaine et de la santé publique et de prendre nos responsabilités pour protéger une ressource essentielle à la vie. Soutenir cette proposition de loi, c'est affirmer le principe universel du droit à l'eau pour tous, autrement dit, du bien commun. Alors, passons à l'acte ! Ce droit nous concerne tous. Nous voterons cette proposition

et à l'assainissement pour les populations les plus fragilisées, comme l'exige la récente directive européenne sur l'eau. L'accès à l'eau et la protection de cette ressource sont l'un des défis majeurs de notre siècle. L'eau est à ce point essentielle qu'elle conditionne tout simplement c'est le cas de l'ensemble des biens communs, les politiques de marchandisation et de libéralisation ont conduit à rendre son accès plus difficile et plus onéreux.

La perte d'ingénierie publique tout comme les regroupements XXL ont poussé les collectivités à déléguer cette compétence, livrant les usagers aux mains des opérateurs privés comme Suez ou Veolia. Face à cette situation, cette proposition de loi pose un principe simple : si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit universel, alors, pour la proportion qui est vitale, cet accès doit être gratuit pour toutes et tous et sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une exigence d'égalité et de solidarité qui découle de nos engagements internationaux tout comme de l'article 1 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. est la responsabilité des pouvoirs publics qui, lorsqu'ils reconnaissent un droit constitutionnellement ou législativement, doivent parallèlement créer les conditions de son effectivité. Alors que selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté 1 million de Français, qui s'ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté, nous souhaitons, à l'image de l'exigence exprimée par les « gilets jaunes », allier performances écologiques et exigence de justice sociale. Il n'y aura pas de transition écologique réussie sans partage des richesses, du savoir et des pouvoirs. Nous allions donc concrètement protection des biens communs et accès aux droits, en l'occurrence, au droit à l'eau. Certains nous répondent que nous avons déjà fait beaucoup en interdisant les coupures. C'est un premier pas, mais un droit ne se définit jamais par la négative. Permettez-moi de revenir sur deux points qui nous paraissent importants. Au-delà de sa dimension sociale, cette proposition de loi pose une question plus générale, celle de la gestion d'un bien commun.

Pourtant, chers collègues, il faut également entendre l'exigence qui s'exprime dans beaucoup de territoires pour le retour aux régies. Cela s'explique simplement par le constat que, pour protéger les biens communs, les services publics sont bien les outils les plus pertinents et performants. Par ailleurs, comment ne pas penser aux tentatives monopolistiques en cours entre Suez et Veolia et à leurs conséquences sur les usagers de l'eau, considérés comme de simples réservoirs de profits à venir ? Les pouvoirs publics doivent intervenir pour sortir l'eau de ces politiques de marchandisation à rebours des exigences

Enfin, nous ne nous félicitons pas de l'OPA hostile de Veolia sur Suez. Il ne s'agit pas d'un accord, mais bien d'une capitulation qui aura des effets graves sur le long terme pour les collectivités, les usagers et les salariés. Il est urgent de constituer un grand service public national de l'eau par la création d'un pôle public réunissant tous les acteurs économiques et garantissant l'égalité du prix de l'eau et l'accès à tous partout sur le territoire national. Cela permettrait de fédérer les acteurs publics aujourd'hui dispersés, coordonner les investissements publics et privés indispensables et de faire converger les compétences et les savoir-faire. Cet outil au service de la maîtrise publique de l'eau doit permettre une gestion démocratique associant les usagers, les collectivités et tous les acteurs de la filière. la filière. Il s'agit enfin d'une condition indispensable à la défense de l'emploi et des savoir-faire, mais aussi d'un levier indispensable pour garantir une gestion de cette ressource

je remercie l'auteur de la proposition de loi et le rapporteur pour leur travail sur ce texte, qui est directement inspiré de la proposition de loi visant à la mise en oeuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement examinée, puis rejetée par le Sénat le 22 février 2017. Ces deux textes sont l'aboutissement de travaux menés en lien avec des associations et ONG afin de rendre effectif le droit d'accès à l'eau en permettant que les personnes les plus vulnérables disposent d'un accès aux équipements sanitaires indispensables et de mettre en place une aide préventive pour l'eau. L'objectif est évidemment louable : l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental inscrit dans plusieurs traités internationaux. Le droit à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène constitue notamment l'objectif n° 6 des dix-sept objectifs de de développement durable 2030 adoptés par les États membres des Nations unies qui visent à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et à un assainissement gérés de façon durable. C'est une question de salubrité, d'hygiène et de santé publique. Le Sénat avait cependant été conduit à rejeter le texte de 2017 pour de multiples raisons. D'abord, parce que celui-ci introduisait des obligations nouvelles pour les collectivités territoriales à l'article 2, notamment l'installation d'équipements de distribution gratuite d'eau potable, de toilettes, de douches publiques et de laveries gratuites. Ensuite, parce que les articles 3 et 4 introduisaient deux aides préventives pour l'accès à l'eau en sus des aides curatives, en utilisant le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées, dont les sommes perçues par la douane sont mises à la disposition de chaque commune concernée. examinons aujourd'hui reprend très exactement les dispositions de la proposition de loi précitée. Il remplace néanmoins les deux mécanismes financiers qu'elle prévoyait par un principe de gratuité des premiers mètres cubes d'eau. En commission, le rapport a été rejeté au motif que le dispositif introduit des obligations nouvelles pour les collectivités territoriales et que, en l'absence d'étude d'impact, il est impossible de chiffrer le coût de cette mesure- coût de mise aux normes, d'entretien et coûts d'acquisition de locaux dédiés. La question que nous pourrions nous poser est la suivante : quelles sont les solutions opérationnelles que nous pouvons apporter pour permettre à tous l'accès à l'eau dans des conditions économiques raisonnables, aussi bien pour les usagers que pour les collectivités La gratuité de l'accès à l'eau pose problème. En effet, il est d'autant plus nécessaire de préserver les ressources que, dans un contexte de dérèglement climatique, l'eau est et sera de plus en plus rare. Une vigilance s'impose ; or sobriété ne rime pas avec gratuité. Il est de notre responsabilité de trouver un mécanisme de solidarité qui ne mette pas à mal le modèle économique de l'eau, notamment en exerçant une pression financière sur les collectivités.

À moyen terme, il faudra sécuriser les budgets, et même les rehausser de plusieurs milliards d'euros afin de parvenir à un niveau d'investissement à la hauteur des besoins de renouvellement de nos réseaux, de faire face à l'adaptation au changement climatique et d'accompagner nos collectivités dans ces évolutions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je commencerai mon intervention par une remarque bienveillante à l'endroit de nos collègues du groupe CRCE.

Malheureusement, ces progrès ne suffiront pas pour orienter le groupe Les Républicains vers un vote favorable ou même une abstention. J'ai parlé de « progrès », car cette proposition de loi a été expurgée des deux dispositions du texte de 2017 que nous avions combattues avec vigueur l'aide préventive pour l'eau, prévue à l'article 3, et la création d'une allocation forfaitaire d'eau pour les ménages les plus pauvres, lorsque le prix de l'eau dépasse un prix de référence fixé par décret, à l'article 4.

surtout hostiles au fait que l'allocation soit issue du produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées, dont les sommes perçues par les douanes sont mises à la disposition de chaque commune concernée. Où est le problème dans le texte dont nous débattons aujourd'hui ?

et, surtout, en l'absence d'étude d'impact, il est impossible d'en chiffrer le coût, qu'il s'agisse du coût des mises aux normes, du coût d'entretien ou du coût de l'acquisition des locaux dédiés. S'agissant de l'article 3, le principe de gratuité des premiers mètres cubes me semble plus simple à mettre en place que les allocations prévues par le texte de 2017. Je pense, néanmoins, qu'il ne faut pas poursuivre dans cette direction, si l'on veut éviter de voir se multiplier des principes de gratuité injustifiés. en effet, déjà, chaque année, dans l'obligation d'écraser des centaines de milliers d'euros de factures impayées. Vous l'aurez compris, malgré un objectif louable, je voterai contre cette proposition de loi. J'ajouterai deux remarques pour justifier ce rejet. d'abord, je considère qu'il existe d'autres priorités en matière d'infrastructures. La gestion de l'eau nécessite, en effet, des investissements massifs dans les infrastructures d'alimentation en eau, car leur rythme actuel de renouvellement est de deux cents ans ! Avant de réaliser des infrastructures ou des installations dont on ignore si elles seront utilisées, il faudrait plutôt agir sur les réseaux fuyards et, surtout, remédier au désengagement croissant de l'Agence de l'eau, qui finit par faire tout autre chose que ce pour quoi elle a été créée.

encore amplifier les aides sociales. Nous oublions trop souvent que les situations de détresse sociale ne tombent pas du ciel et que nous avons les moyens de les combattre en amont. Avant le droit individuel à l'eau potable, je crois qu'il y a un droit pour la France, donc un droit collectif, à avoir une agriculture de nouveau puissante et une industrie de nouveau florissante, pour que nos compatriotes retrouvent l'emploi qui les préserverait de telles situations de détresse. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Je mets aux voix l'article 1.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements, ma compassion et mon soutien aux associations qui défendent ce droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Nous restons mobilisés pour faire valoir ce droit fondamental et inaliénable.